La séance est reprise. Monsieur le 1er ministre et messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité ou de gouvernement et sont retransmises en Direct sur France 3 et Public Sénat sur notre site, chacun sera attentif au respect des uns des autres et autant de parole et nous commençons par notre collègue Alain Fouché pour le groupe, les indépendants pour 2 minutes chers collègues. Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, ma question porte sur la protection des propriétaires et locataires contre les professionnels du squat, la presse fait régulièrement écho de propriétaires et locataires qui après s'être absenté de leur domicile principal pour les vacances ou un simple week-end, le retrouve occupé par des squatters, ces professionnels du squat investissent les lieux change les serrures et imposent leurs noms sur la boîte aux lettres, il ne s'agit pas de locataires qui ne paient pas leur loyer, mais d'individus qui commettent un délit pénal réprimé par l'article 226 4 du code pénal passible d'un an de prison et de 15000 euros d'amende si la loi Dalo de 2007, a créé un droit au logement garanti par l'État, elle a en contrepartie créer une procédure administrative d'évacuation forcée en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, cette procédure permet à une personne à tout moment de faire évacuer de son domicile principal les squatter sans intervention du juge ni application du délai de flagrance de 48 heures dans les fêtes, cette procédure ne reçoit que peu voire aucune exécution aussi, monsieur le ministre d'État, je retour et savoir quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour garantir l'effectivité des droits des propriétaires et des locataires. Pour vous répondent : la parole et avec Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, monsieur le ministre, pour 2 minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je vous remercie de de votre question parce que ça va me permettre de rappeler très clairement effectivement quel est le droit aujourd'hui, qui plus est dans un contexte où ces dernières heures, ces derniers jours, nous avons pu lire ici ou là des informations qui étaient fausses, votre question, Monsieur le Sénateur, porte sur la protection du domicile dit principal le lieu d'habitation, contrairement à ce que nous avons pu lire la loi la sécurité juridique aujourd'hui est forte vis-à-vis de ces squatters qui peuvent venir occuper votre domiciliation principal quelles sont ces sécurités il y a d'abord la loi Dalo que vous avez mentionné cette fois de 2007, qui permet effectivement une procédure administrative, par le truchement du préfet, le préfet qui à ce moment-là peut saisir soit les je dirais juridiction soit la police compétente mais surtout à partir de 2015 à partir de la loi du 24 juin 2015, il a été reconnu que l'infraction porté non seulement sur l'entrée dans les lieux, mais également sur l'occupation illicite de ces lieux, c'est-à-dire de du domicile principal de l'occupant et cette fois, de juin 2015 permet désormais à la police d'intervenir au titre de la flagrance pour déloger les squatters qui se trouvent dans ces lieux et ce qui est important de préciser, c'est que ce fameux délai de 48 heures ne s'applique aucunement, aucunement au regard de cette loi et donc vous avez raison, Monsieur le Sénateur, il y a aujourd'hui également un problème de communication vis-à-vis des procédures vis-à-vis du droit existant, si demain quelconque aperçoit des squatters venir prendre pied dans votre résidence principale, il faut prévenir la police, la police depuis juin 2015, alors la nécessité la nécessité d'intervenir au titre de la flagrance et le fait de communiquer dessus, permettre à chacun de rappeler les responsabilités qui sont les leur je vous remercie. J'ai déposé une proposition de loi cosignée par de nombreux collègues que je remercie qui tend à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale, lorsque les squatters occupent le domicile principal dans les fêtes, les personnes s'adressent aux services de police qui souvent refusent d'intervenir, donc il est bon de faire passer une circulaire, le locataire ou le propriétaire est alors obligé de prendre un avocat et de saisir le juge pour qu'il ordonne l'expulsion du squat, voire la suppression de la trêve dire cette procédure dure des mois, donc je compte sur vous Monsieur le Ministre, pour soutenir la proposition de loi quand elle sera déposée. La parole est à notre collègue a une marcher pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale Monsieur le Ministre, aujourd'hui, le monde rural rime trop souvent avec l'abandon enclavement déserts médicaux zones blanches numérique fermetures de commerces, disparition des services publics, nous apprenons que pour la rentrée prochaine, c'est au tour des écoles rurales d'être sacrifiés décision couperet sans aucune concertation avec les élus locaux, alors que ceux-ci entreprennent de construire des écoles qui sont le coeur battant de nos communes, le dédoublement des classes de CP dans les REP et de CE1 dans les raids plus est une bonne chose, mais pas au détriment des classes du monde rural, personne n'est dupe, Monsieur le Ministre et les territoires ruraux en ont assez d'être dépouillé au profit de vos politiques publiques, c'est un aveu de mépris et de plus, là où la scolarisation des enfants méritent autant de moyens que partout ailleurs, de toute la France, les nouvelles de menaces de fermeture de classe en milieu rural se répandent des exemples, 84 dans le Pas-de-Calais 51 dans l'Oise 46 en Meurthe-et-Moselle 27 en Moselle 66 dans les Vosges 15 en Corrèze 45 en Eure-et-Loir 121 en Seine-et-Marne, mon département dont parfois plusieurs dans une même commune comme à soupe sur loin alors que peu d'ouverture sont annoncés pourquoi votre gouvernement accorde-t-il tant d'attention aux enfants et si peu aux autres comment expliquez-vous cela, monsieur le Ministre, les petits écoliers Deschamps ne serait-il pas égaux en droits à ceux des villes. Pour vous répondre, la parole est à monsieur ministre de l'éducation. Nationale Jean-Michel Blanquer. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices madame la sénatrice merci pour votre question qui me permet de préciser ce sujet d'équilibre entre l'urbain et le rural, mais je voudrais d'abord et avant tout dire à quel point il n'y a pas en ce moment de sacrifice du rural au profit de l'urbain, ça n'est pas exact, je vais le dire avec des chiffres, il y a plus de 30000 élèves en moins l'année prochaine dans les écoles primaires de France nous créons 3800 postes dans chaque département rural de France et je m'engage en le disant, il y aura plus de professeur par élève à la rentrée prochaine, ce n'est pas tout à fait honnête de citer les fermetures de classes dans chacun des départements, comme vous l'avez fait en ne mentionnant pas les ouvertures en ne mentionnant pas les ouvertures dans le même département, je prends votre département, Madame la sénatrice, la Seine-et-Marne, que je connais bien et que vous avez cité il y a 240 élèves en moins à la rentrée prochaine, il y a 40 professeurs supplémentaires dans votre département et il y a dans votre département, 30 dédoublement à la rentrée dernière, 70 à la rentrée prochaine, donc la Seine-et-Marne bénéficient de cette mesure, comme beaucoup, départements, y compris parfois en milieu rural et votre département non seulement n'aura pas un taux dégradée mais aura un taux augmenter alors je vois bien qu'on essaye d'installer une petite musique pour essayer un petit peu de dénigrer la mesure de dédoublement, mais le gouvernement s'est donné les moyens de faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire le dédoublement en zone urbaine, mais aussi parfois en zone rurale et une politique rurale volontariste à laquelle je vous invite à vous associer, donc nous n'avons pas avoir des analyses fausses nous avons avoir des analyses conjointes et ensuite faire en effet renaître le rural grâce à l'école, je suis engagé par une politique d'attractivité des territoires ruraux, notamment par les contrats département auquel je travaille d'ailleurs avec Jacques Mézard pour que justement, nous ayons une renaissance du rural, merci à vous. Nous savons que la réussite de nos jeunes se joue dès la maternelle et l'école élémentaire, l'État doit mettre toutes les chances du côté de tous ces écoliers sans discrimination lors de la conférence des territoires du 17 juillet dernier : le président de la République a affirmé pompeusement que les territoires ruraux ne peuvent plus être la variable d'ajustement et qu'il n'y aura plus aucune fermeture des places dans les écoles rurales, bonsoir Monsieur le Ministre, comment pouvez vous répond de la sorte, vous qui avez été un recteur d'académie appréciée des élus que j'étais et qui connaissait les difficultés du monde rural, écoutez, écoutez bien Monsieur le Ministre,

La parole est à notre collègue Pierre eau pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, Monsieur le 1er Ministre Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le même sujet mais c'est là un sujet d'importance pour les territoires ruraux, je crois que ça n'est pas affaibli, on est sur une période où 75 pourcent de notre territoire est en cours d'abandon par l'État par les services publics et je crois que les fermetures d'écoles et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on parle d'aider les zones d'éducation prioritaire, est-ce que des territoires ruraux, où un enseignant à 3, 4, 5 niveaux différents dans une même classe est-il logique d'appliquer les mêmes normes de 25 voiles appauvrir pour fermer une classe, ce sont des normes de 25 à la ville comme à la campagne, je pense qu'il faut réduire cette norme pour les territoires ruraux et la ramener à 20 20 permettrait effectivement de prendre en compte cette difficulté des enseignants ruraux, il y a un 2ème point que je tiens à souligner, c'est la longueur des déplacements, j'ai bien compris qu'il fallait être volontaire pour réorganiser les classes sur les territoires ruraux mais on a créé des regroupements scolaires 3 ans après on ferme une classe quand on ferme une quand on ferme une école parce qu'il y avait 2 classes dans une école et à nouveau on repart mouton à saute-mouton vers de nouvelles réformes je crois véritablement, monsieur le ministre, qu'il faut prendre conscience de cette difficulté des territoires ruraux, je demande également au 1er ministre de prendre en compte toutes les problématiques, on le voit bien les manifestations pour les problèmes de zonage européen. On fait ça vu de Paris, conclut avec des normes qui échappent véritablement au territoire. monsieur le sénateur, je je me permet d'aller vite, puisque c'est la même question que tout à l'heure, et donc elle me permet de prolonger le propos mais je commencerai par là où j'ai fini tout à l'heure, c'est-à-dire je vais parler de votre département, parce que comme ça, chacun verra que pour chaque département je peut en effet dire la même chose, c'est-à-dire que le taux d'encadrement s'améliorer en ce qui me concerne c'est l'Indre-et-Loire dans le 1er degré, il y a 104 élèves en moins l'année prochaine pour autant, il y a 12 postes qui sont fléchés pour les dédoublements en REP 12 postes qui sont fléchés pour le remplacement et 16 postes qui sont fléchés pour soutenir les écoles rurales, concrètement, il y a 6 postes supplémentaires alors qu'il y a moins d'élèves, il y a donc vous le voyez, une réalité cette réalité, elle sera vrai pour chaque département et je suis disponible pour tous les représentants de chaque département rural de France pour en parler concrètement, je crois que nous avons un point d'accord et un point de désaccord, le point d'accord, il est évidemment celui de la nécessité de la renaissance du monde rural et vous ne trouverez toujours à vos côtés pour cela et nous y travaillons en ce moment, nous y travaillons donc au travers des contrats ruraux de départements, j'y faisais référence tout à l'heure avec Jacques Mézard, c'est un point très important puisque, en ce moment même, nous invitons les départements qui n'en ont pas aller signer à chaque fois que nous les c'est 5 postes supplémentaires que nous donnons pour la renaissance du rural, nous devons avoir des stratégies partager pour sauver les écoles et même mieux, pour les rendre plus attractives, vous avez parlé des classes multiniveaux les classes multiniveaux, c'est en effet en fait un atout pédagogique, c'est grâce aux classes multiniveaux que les écoles primaires rural ont de meilleurs résultats que les écoles primaires moyenne en France, donc je suis pour des écoles primaires rural tonique, nous devons les faire renaître, nous sommes en train de nous en donner les moyens et là où nous avons un petit point désaccord bien moins important que notre point d'accord, c'est que je pense qu'il ne faut pas tenir de discours de déploration au moment même où il y a un travail de renaissance, nous devons être tous associer pour ce travail de renaissance, nous nous en sommes donnés les moyens, ce sont des choix budgétaires très importants si nous répondons si nous accentuant désespoir dans la population par des discours qui ne correspondent pas à nos priorités, nous nous faisons du tort, mais si nous travaillons ensemble à cette renaissance, nous y arriverons, et en tout cas c'est l'invitation que je vous fais, je suis disponible pour tous les représentants, département par département pour une stratégie de renaissance du monde rural, merci. la parole est au président François Patriat pour le groupe, la République en marche, vous avez le président. ça Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est de Bretons donne aux questions d'actualité de faire part au gouvernement de sujets d'inquiétude de de difficultés dans notre pays, moi je voudrais poser une question de gouvernement sur un sujet d'actualité qui intéresse tous les Français, c'est celui aujourd'hui de la valeur travail et du redressement de notre économie. Ce matin, l'INSEE a publié les chiffres concernant le chômage. Chers Chers collègues, je suis très heureux de voir que l'amélioration du chômage suscite des cris d'orfraie dans cette hémicycle je salue ici l'engagement de tous les parlementaires qui participent au redressement de notre pays, mais enfin en publiant ce matin, le fait qu'il y a 200 ça 1000 chômeurs de moins dans notre pays, que le taux de chômage en France métropolitaine, soit de 8 6, 8, 9 tout territoire français on montre que les efforts qu'ont menée les uns et les autres, beaucoup de ces armées ont porté leurs fruits et je voudrais poser ma question à la fois sans triomphalisme avec objectivité en disant qu'à la fois la croissance à la fois des décisions prises antérieurement mais surtout des décisions prises par ce gouvernement pour redonner la confiance, ont permis de créer un climat dans ce pays un climat et une dynamique qui va dans le redressement, je sais que les mesures de simplification, les mesures pour l'apprentissage, les mesures pour la formation des mesures qui aujourd'hui permettent à la fois au salarié aux entreprises de trouver plus de liberté, de conduire alors ma question que c'était pas cher collègue ma question au gouvernement de dire monsieur le 1er ministre, pensez-vous que cette pente qui aujourd'hui s'accentue, est un signe qui pourra se poursuivent et, à ce que les décisions futures du gouvernement avec les 10 chantiers mis chers collègues, nous allons avoir à traiter, a voté ici permettront cette embellie se poursuive, je vous remercie, qu'il vous plaît, monsieur le 1er ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Patriat. Je n'ai pas beaucoup de doute que si les chiffres qui avaient été publiées ce matin, n'avait pas indiqué la diminution au cours du dernier trimestre. Du chômage à hauteur de 250000 emplois, je n'ai pas beaucoup de doute sur le fait que tout le monde ici aurait pris les statistiques au sérieux et sur le fait que beaucoup en aurait tenu responsable le gouvernement. reconnaissez-le. Il se trouve, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'en effet, il se trouve qu'en effet ce matin l'INSEE a publié les chiffres du chômage : les chiffres trimestriels car vous avez peut-être remarqué, mesdames et messieurs les sénateurs, que le gouvernement a décidé de s'abstenir de commenter les chiffres mensuels pour rester sur le commentaire et l'analyse des chiffres trimestriels qui sont faits par l'INSEE au sens du Bureau international du travail, et qui sont plus robustes dans leur présentation et dans leur définition que les simples chiffres mensuels que montrent ces chiffres que le taux de chômage en France s'établit, au moment où nous parlons, à 8,9 pourcent de la population active, c'est son plus bas niveau depuis 2009. Est-ce que je m'en réjouis, avant de vous réponde, je voudrais quand même vous dire à quoi correspondent 8,9 pourcent de la population active, c'est très exactement, mesdames et messieurs, 3 1000000 709500 personnes qui sont au chômage en France le 1er qui osent se réjouir. Doit être mis face à face avec ce chiffre, il y a encore dans notre pays 3 1000000 700000 chômeurs, le chiffre s'améliore tant mieux 2ème chiffre qui s'améliore et c'était là aussi, tant mieux, le taux d'emploi dans notre pays, c'est un indicateur important, le taux d'emploi était en descendant de 65,7 pourcent il est supérieur à tous les autres chiffres en la matière depuis le début des années 80 est-ce qu'on peut s'en réjouir, oui, bien sûr, est-ce que le travail est fini, non, bien entendu et je voudrais dire, mesdames et messieurs, que nous voulons, en la matière, non pas célébrer une victoire, une petite victoire, une victoire quand même la victoire a toujours 1000 pères. Nous voulons gagner une bataille et une guerre durablement nous voulons gagner la bataille contre le chômage de masse et pour gagner ce pour pour remporter cette bataille durablement nous devons attaquer le problème par tous les bouts, c'est ce que nous avons commencé à faire sans renier rien de ce qui avait pu être fait auparavant, quelles que soient les gouvernements, mais en essayant d'apporter des réponses durables, car il nous semble que le problème est depuis trop longtemps, enracinée dans la réalité économique française, cela veut dire effectivement, comme nous l'avons fait et je voudrais remercier le Sénat modifier le code du travail lorsqu'ils constituent quelque chose qui nous paraît de nature à freiner les embauches dans notre pays, cela veut dire transformer la fiscalité Kant la fiscalité nous paraît de nature à freiner les embauches dans notre pays, cela veut dire transformés et améliorés et, ô combien, améliorer le système de formation pour que, depuis l'école primaire, le ministre de l'Éducation nationale en parler jusqu'à la formation professionnelle en passant par le bac par l'accès à l'enseignement supérieur et par l'apprentissage nous puissions élever le niveau de compétence de nos concitoyens car c'est par l'élévation du niveau de compétences que l'on peut réduire durablement le chômage, tout le monde le sait, tout le monde se bat pour que ses propres enfants acquièrent le le meilleur niveau de compétences possible parce que tout le monde sait que c'est la meilleure sécurité contre le chômage, nous voulons donc agir massivement dans tous les domaines pour que la France puisse enfin rejoindre l'ensemble des pays qui ont un taux de chômage largement inférieur à celui qui prévoit encore. Merci monsieur le 1er ministre. La parole est maintenant notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le 1er Ministre je voudrais vous parler de sa robe sa couleur brillante de ses effluves parfumées de ce Patrimoine français de cette culture de l'excellence, je voudrais vous parler tout simplement du vin, vous parlez de nous les vignerons de la terre que nous avons façonné pendant des siècles pour en faire des terroirs de renom de nous, chefs d'entreprise qui créeront des emplois malgré grêle Cégétel et qui faisons notre révolution environnementale, qu'elle soit bio ou achever eux car nous sommes avant tout des femmes et des hommes responsables le vin se boit avec modération mais extase et ne saurait être ramenée à la seule dimension d'une boisson contenant de l'alcool, la profession ne saurait être pointés du doigt, alors que nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur une politique de consommation responsable le candidat Macron un verre à la main et annoncé que la viticulture était une part vibrante de nos territoires et je rajouterai une part importante de notre économie, 10 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires à l'export en 2016 le 2ème poste excédentaire de la balance commerciale française par courrier du 19 janvier dernier le président de la République, exprimé son souhait que les acteurs de santé, mais aussi les acteurs économiques que nous sommes s'empare du sujet afin de mener la révolution de la prévention pourtant parallèlement à cette écrit votre ministre de la Santé ne cessent de jeter l'opprobre sur nos têtes, sa stratégie nationale de santé, soit de passer d'une politique de prévention des risques à une politique de prévention de toute consommation d'alcool, mais la consommation de vin a déjà été divisé par 2 en 50 ans sans régler pour autant le problème de l'alcoolisme, cette voie n'est donc pas la bonne, alors Monsieur le 1er Ministre ma question est simple : allez-vous reconnaître les histoires d'une consommation responsable vous souhaitez vous suit votre ministre de La Fontaine, qui veut faire de la France, le pays de la prohibition allez-vous nous précipiter dans un grand plan de licenciements et de démembrement ou allez-, vous décidez de nous associer à notre destin, comme nous l'avons toujours fait

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs Madame la ces détresses permettez à un élu normand. Donc élu d'une région où la production viticole et il faut le reconnaître. Moins importante que dans l'excellence des autres productions agricoles de la région de vous répondent. Comme le président de la République, comme vous, manifestement, comme des millions de Français, j'aime le vin. ça ça n'a pas toujours été le cas, y compris parmi les grands élus de notre pays. pays. Reconnaissez avec moi madame la sénatrice, que l'on peut même sans goûter aux produits reconnaître l'importance de ce qu'est le vin. La culture de la vigne, l'attachement des Français à ce produit, donc nous pouvons sans conteste, dire qu'il occupe une place particulière dans l'imaginaire et la culture française. Vous nous dites, madame la sénatrice, que le gouvernement par la voix de Madame la ministre des solidarités, de la santé seraient engagés dans je ne sais quelle croisade contre le vent. Permettez-moi de vous dire madame la sénatrice que votre propos que j'entends, je respecte ma apparaît, pardon pour ce terme outrancier. Je le dis comme je le pense, pourquoi d'où tirez-vous madame la sénatrice que ce gouvernement aurait pris des mesures défavorables aux viticulteurs et à la culture du vin en général, si je puis dire, pas dans les négociations internationales que nous menons, qui sont menés en ce moment par la Commission européenne et dont vous savez madame la sénatrice même si peu de gens le disent qu'ils permettent des exportations plus aisés et des protections plus solide pour les producteurs français, je me sers madame la sénatrice que souvent on dénonce c'est ces négociations commerciales en oubliant, y compris ceux qui font démonstration d'amour et de défense de la profession viticole que c'est négociations ont souvent pour objet ont souvent pour effet de permettre l'exportation a crû et dans de meilleures conditions, des produits français, avez-vous vu madame la sénatrice que ce gouvernement et modifier en quoi que ce soit la fiscalité applicable au vin, il n'en est rien, si vous pensez, Madame la sénatrice qu'une ministre des solidarités et de la santé qui, toute sa vie professionnelle a été médecin, professeur d'hématologie va dire publiquement. Que le vin ne comporte pas d'alcool et que l'alcool peut avoir peut avoir un impact dans des questions de santé publique. Si vous imaginer cela une seconde, c'est que vous ne comprenez pas, je le crains, ce que nous souhaitons faire respecter, respecter et développer développer une pratique modérée, je crois que tout le monde ici accepte l'idée qu'il faille boire le vin avec modération, alors de grâce. non mais franchement, si vous considérez qu'il y a pas de sujets de santé publique, on peut en parler. C'est pas le 20. Eh bien nous, madame la sénatrice, ce que je vous propose, c'est que nous allons regarder le problème en face et que nous allons à la fois respecter cette place particulière à laquelle nous sommes tous attachés du vin dans l'activité et dans l'agriculture française, mais que nous n'allons pas faire semblant qu'il n'y aurait pas de problème de santé publique, parce qu'il y aurait quelque chose de profondément irresponsable à ne pas voir les 2 faces de la même pièce. La parole est maintenant notre collègue Dominique votre pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologistes 2 minutes chacun respecte son temps. Madame la ministre de la santé, bonne, il n'y aurait pas le ras-le-bol des professionnels de santé qui s'exprime dans les luttes en cours et que les parlementaires communistes entendent aussi dans le cas du Tour de France des hôpitaux et des Epad qu'ils viennent d'engager oui, notre système de soins se dégrade et vite, oui, le temps des rafistolages est révolu, ce n'est pas non plus nous qui vous contrediront sur les exigences de prévention, ce qui pose aussi la question de la santé au travail que les gouvernements successifs ont mis à mal, ou la nécessité de réévaluer les formations médicales, mais encore faudrait-il donner aux universités les capacités d'accueil, une réforme d'ensemble, oui, mais quelle réforme et avec quels moyens depuis 10 ans se sont moins 7 milliards d'économies à marche forcée qui ont été imposées à l'hôpital public, au moins 1,4 milliard dans votre seul budget de la Sécurité sociale pour 2018 plus 2 virgule 3 pourcent de progression alors que les besoins sont estimés à plus 4 dans ces conditions, l'enveloppe annoncée de 100 millions d'euros en même temps qu'une nouvelle ponction sur les tarifs à l'activité est vécue comme une aumône, voire une insulte par le monde médical et les personnels soignants confrontés ou toujours faire plus avec toujours moins nous disons chiche à votre annonce de concertation, nous ne manquons pas de propositions pour construire ou reconstruire un service public territorialisée coordonnées de santé avec tous les acteurs de santé le concerné plutôt que de déréguler le droit du travail à l'hôpital public ou mettre le privé sur le même plan que le public, comme vous l'annoncez la finance n'a déjà que trop de place à l'hôpital, à l'hôpital public déjà terriblement endetté par les politiques d'austérité, Madame la Ministre, accepterez-vous de rencontrer les parlementaires communistes pour réentendre, à l'issue de ce Tour de France, et avant d'annoncer votre plan les témoignages et propositions recueillies, notamment celle d'un plan d'urgence pour les hôpitaux. Vous répondent : la parole et. Madame la ministre des solidarités, de la santé pour 2 minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vatrin d'abord bien entendu je vous rencontrerai, bien entendu, car cette concertation doit concerne évidemment tous les citoyens, les élus, les professionnels, mais les élus de territoires sont les premiers concernés par les modifications aujourd'hui du système de santé et la difficulté d'accéder à des soins de qualité, alors vous l'avez dit, la situation financière des hôpitaux s'est beaucoup dégradée devrait aujourd'hui friser le milliard de déficit déficit consolidé en 2017, c'est donc un doublement par rapport à l'année précédente et c'est lié à une stagnation de l'activité des hôpitaux, la régulation de nos dépenses de santé aujourd'hui qui est fondée sur l'activité des des établissements de santé ne permet pas d'amortir les diminutions d'activité, le virage ambulatoire, il nous faut donc donner des leviers aujourd'hui aux établissements pour adapter leur rôle aux évolutions des besoins, notamment face à l'émergence de maladies chroniques, face aux besoins de prévention face à la difficulté de trouver un médecin dans des épaves par exemple, pour cela, le 1er ministre l'a annoncé : nous avons décidé d'une transformation globale et cohérente de notre système de santé et nous débutons une concertation, nous allons essayer de mieux articuler la médecine de ville et la médecine hospitalière avec des tarifications parcours de soins, développer des organisations innovantes, incluant le médico-social, vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, le temps des rafistolages est révolu, nous lançons 5 chantiers de concertation sur les organisations territoriales sur les ressources humaines sur le numérique sur la tarification sur la pertinence des actes tous les citoyens de ce pays seront amenés à donner leur avis sur une plateforme en ligne en dehors évidemment des concertations territoriales que nous débutons à la fin du mois, je vous remercie. Merci madame la ministre, la parole est maintenant notre collègue Jean-Luc ici pour le groupe socialiste et républicain. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des solidarités et de la santé, madame la ministre, vous avez rendu public ce mardi, avec le 1er ministre aux ambitions en matière d'organisation des soins dans notre pays, ce n'est pas nouveau notre pital public souffrent nos concitoyens ont du mal à trouver une offre de soins cohérente depuis 2009, de nombreux dispositifs ont été mis en place, pourtant, les médecins sont de plus en plus absent de nos territoires et la population est de plus en plus inquiète, vous souhaitez une meilleure cohérence entre l'hôpital et la médecine générale dans l'objectif de placer le patient au coeur du dispositif de soin, nous le souhaitons également, mais nous ne voyons pas dans vos annonces, ce qui pourrait permettre l'installation de médecins généralistes, là où il en manque, l'État et les collectivités locales, financer l'installation des médecins sans résultat probant aussi nous semblerait-il judicieux de rendre public l'ensemble des financements locaux et nationaux en matière d'installation des médecins pour en aux jurés l'impact, êtes-vous prêt à faire ce bilan Madame la Ministre, par ailleurs, les Groupements hospitaliers les territoires j'acheté vise à mutualiser l'offre hospitalière sur un territoire donné, or on constate le plus souvent une stratégie d'offre de soins très concentré sur le plus grand établissement hospitalier au détriment des plus petits, la réponse en la matière ne saurait être la télémédecine comme l'Alpha et l'oméga de l'offre de soin dans les déserts médicaux sur ces 2 points, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions, je vous remercie. Bon vous répondent cette fois-ci, la parole est à la ministre des solidarités, de la santé avait la parole. évidemment, nous sommes prêts à rendre publics tous les financements incitatifs qui ont été proposées par les uns et par les autres, nous sommes prêts évidemment faire ce bilan mais nous pensons, comme vous, quelque part, que les mesures incitatives ne suffisent pas, aujourd'hui, face à la difficulté que rencontrent les territoires, nous avons avec le 1er ministre dès le mois d'octobre, proposer un plan dédié à l'accessibilité aux soins qui mise sur 3 changement de paradigme, le 1er c'est qu'un médecin n'a pas forcément besoin de s'installer dans un territoire il faut donner à chaque territoire du temps médical et ce temps médical peut venir de l'hôpital de d'autres professionnels de de santé hospitaliers et chaque territoire doit trouver les leviers pour favoriser cette projection de temps médical sur un territoire sous-dotées, le 2ème changement de paradigme, ce sont les coopérations inter-professionnel, c'est aussi un changement culturel, toutes les maladies non pas besoin systématiquement d'être suivis par un médecin, un patient qui je souffre d'une hypertension artérielle aujourd'hui peut être suivie par une infirmière, à condition que ces soins coordonnés s'inscrivent dans des coopérations réguler et ce que font aujourd'hui la plupart des maisons de santé pluri-professionnelle le 3ème changement de paradigme, c'est la télémédecine, bien sûr, ce n'est pas l'Alpha et l'oméga mais ça peut ralentir raccourcir Des délais de prise en charge, l'autre changement de paradigme, c'est aussi le fait que nous faisons confiance aux territoires, nous leur donnons 26 leviers d'action 26 mesures qui leur permette de d'adapter leur organisation territoriale, avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de liberté aux besoins de chaque territoire nous dédions 400 millions d'euros dans le grand plan d'investissement à la création de maisons de santé pluri-professionnelle dont nous souhaitons doubler le nombre d'ici la fin du quinquennat mais ça aussi, ça n'est pas l'Alpha l'Alpha et l'oméga de la médecine de demain et donc c'est 26 mesures, elles sont à la disposition des territoires, les ARS vont animer en région dans chaque territoire des réflexions avec les élus, les professionnels de santé, les citoyens pour trouver la réponse la plus proche, plus appropriée pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, je vous remercie.

de dire que l'incitatif de suffit plus et je pense qu'il faudra se poser réellement la question du commerce il tifs vis-à-vis des professionnels de santé, sinon nos territoires resteront dépourvues d'offre et de médecins généralistes, merci. merci. La parole est à notre collègue Jean-Marc Boyer pour le groupe, les républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports, madame la ministre, un espoir a pu naître concernant les transports ferroviaires et le TGV, lorsque vous affirmez en novembre dernier au Sénat concernant votre loi de programmation des infrastructures, je tiens à vous assurer que les enjeux d'aménagement du territoire seront bien pris en compte et le rapport Duron confirmant premières bord la priorité de réduire les inégalités territoriales en assurant de meilleures accès pour les villes moyennes et les territoires ruraux et quelle déception de découvrir ensuite que nombre de projets de la loi sur le Grenelle de l'environnement sont balayées d'un revers de la main. Aussi le grand centre Auvergne Massif central qui comprend 17 millions d'habitants peut s'asseoir sur sa mobilité ferroviaire et son désenclavement et que dire de Clermont-Ferrand que ce rapport condamne à être la seule capitale régionale la plus éloignée de Paris en temps de transport ferroviaire. avec mon collègue Rémy point trop remarquable, président de l'association TGV grand centre Paris Orléans Clermont Lyon nous partageons donc la même crainte de ne jamais voir la réalisation de ce TGV, d'où ma question, madame la Ministre, quelle est votre conception du maillage ferroviaire national et de désenclavement des territoires. Alors vous répondent : la parole quand Madame Élisabeth dormi chargé du transport minutes. Le président, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Boyer, vous m'interrogez sur la prise en compte de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon, dans le rapport du conseil d'orientation des infrastructures, je voudrais tout d'abord saluer l'énorme travail qui a été réalisé par ce conseil au cours des derniers mois, conseil, dont je rappelle qu'il associe des parlementaires de tous bords et je salue à cet égard, les présidents des sénateurs Cornu et Dagobert, des représentants des régions, des départements, des agglomérations et donc des experts. Ce travail était indispensable, indispensable pour sortir de décennies de promesses non financées, ce sont 36 milliards d'euros de lignes à grande vitesse qui ont été promis dans tout le pays, des mises à niveau de routes nationales qui sont reportées, là encore, depuis 2 des décennies de contrat de plan en contrat de plan, c'est l'entretien et la modernisation de notre réseau ferroviaire qui a été négligée au cours de de ces dernières décennies et c'est pour s'attaquer à l'ensemble de ses impasses que le Conseil Dorian tation des infrastructures propose une vision globale des infrastructures au service de l'ensemble des territoires avec une priorité à l'entretien et la modernisation des réseaux et au transport de la vie quotidienne c'est une vision sincère qui met en évidence les coûts et donc les ressources qu'il nous faudra dégager et je note que c'est exactement la méthode préconisée par la commission des finances de votre assemblée, dans son rapport, dans son rapport de septembre 2016, infrastructures de transport sélectionner rigoureusement et financer durablement, nous allons donc étudier les différents scénarios présentés par le conseil d'orientation des infrastructures et, in fine, et le Parlement, qui aura à se prononcer sur la loi de programmation des infrastructures avec une vision globale, cohérente et sincère des projets que l'on peut réaliser journées. journées. Monsieur Boyer. Merci madame la ministre, mais quand même. C'est quand même très inquiétant lorsque Monsieur durant la semaine dernière a dit au Sénat, il est mieux de phase et des infrastructures que de les repousser toujours plus loin, de ne jamais le faire. Lors de la venue du président de la République en Auvergne, il y a quelques semaines, les élus locaux de toutes sensibilités, élus départementaux, régionaux lui ont remis une motion affirmant la nécessité de ne lignes à grande vitesse aujourd'hui, nous doutons que cet appel soit entendu, vous le savez, l'investissement dans les infrastructures, transports, conditions de développement et l'avenir tous les territoires, madame la ministre, vous préparez une France à 2 vitesses, avec des trains à petite vitesse, et en même temps des trains grande vitesse avec des lois Express rapide et en même temps des campagnes, condamné aux 80 kilomètres avec des territoires de 1er de cordée et en même temps des territoires avec une avec une France en marche avant et en même temps une France en marche arrière, La parole est à notre collègue Denis pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. Monsieur le président, Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ce soir, près de 2000 Parisiens vont vont recenser anonymement les personnes de la capitale, passant la nuit sans aucun abri à l'occasion de la nuit, de solidarité, la vague de froid et les chutes de neige qui se sont abattues sur la France la semaine dernière ont multiplié les problèmes réseaux ferroviaires et trafic aérien perturbé, routes impraticables usager immobilisé ces blocages certes pénibles ne doivent pas occulter la dure réalité vécue par les personnes sans abri, les plus impactés par ces conditions hivernales extrêmes ainsi 32 départements ont activé le plan grand froid afin d'ouvrir de nouvelles places d'hébergement, renforcer les équipes du SAMU social, intensifier les maraudes et allonger les heures d'ouverture des accueils de jour et de nuit, mais combien de personnes oublié, seul face au froid glacial de la rue, combien de personnes non détecté par les maraudes, combien de personnes obligées de retourner à la rue, dès que la température les exclura du plan d'alerte, nous ne connaissons pas ces chiffres mais il en est un qui est insoutenable depuis le 1er janvier 45 personnes sont décédées dans nos rues en France et nous comptions 403 morts en 2017 si ces conditions climatiques exceptionnelles permettent des mesures exceptionnelles et la mise à l'abri de personnes supplémentaires des réponses durables doit peut-être apporter hébergeait un sans abri au coup par coup pour une nuit et le laisser regagner la rue le lendemain n'hésite pas une réponse, me semble-t-il à la hauteur de la détresse de ces personnes en c'est alors Monsieur le ministre de la cohésion des territoires, quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour faire du logement un levier de réinsertion des personnes en difficulté dans quelle mesure le lancement du plan quinquennal pour le logement d'abord va-t-il permet d'honorer la promesse du chef de l'État formulée l'été dernier, je le cite : je ne veux plus d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus théorie je vous remercie. Pour vous répondre, le ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard. il s'agit de drames quotidiens que nous connaissons dans ce pays, comme malheureusement pratiquement aussi dans tous les pays dits développés à l'exception peut-être de quelques pays nordiques, le gouvernement a pris à bras-le-corps cette problématique comme d'autres l'ont fait avant et nous avons essayé depuis ces quelques mois en enclenchant la la période hivernale, dès le 1er novembre et la période de grand froid, que nous avons activé il y a une dizaine de jours, ces 30 137 départements qui sont la période grand froid face à cette difficulté de réponse, une réponse immédiate ou d'ouvrir plein davantage de place, nous l'avons fait en mettant à disposition 10000 places de plus que l'année dernière, c'est-à-dire plus qu'il n'y en a jamais eu ce qui ne doit pas être pour nous tous une satisfaction, c'est la constatation malheureusement de graves difficultés dans ce pays par rapport à la solitude et à la misère, c'est la première réponse, c'est une réponse efficace, même si on peut considérer toujours qu'elle est insuffisante 2ème réponse : logement, d'abord c'est lancé le plan logement d'abord qui permet de faire passer de l'hébergement d'urgence à un logement pérenne et ce sont, c'est le projet que nous lançons en collaboration avec les collectivités locales, puisque nous avons reçu plusieurs dizaines de demandes d'intercommunalité pour travailler avec nous, là-dessus, pour ouvrir au cours de ce quinquennat et nous commençons en 2018 10000 places de pensions de famille supplémentaires 40000 places d'intermédiation locative car c'est comme cela que nous pourrons avancer tous ensemble et puis je rappelle que la collectivité nationale mais déjà 2 milliards d'euros sur cette question de l'hébergement d'urgence, certes, on peut toujours faire plus, sachez en tout cas que nous travaillons au quotidien parce que c'est vraiment un drame humain qui nous regarde tous. Merci monsieur ministre. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe, la République en marche la parole pour 2 minutes chacun respecte son temps. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé, Madame la Ministre, le gouvernement a annoncé récemment une refonte audacieuse et globale ayant pour objectif d'optimiser l'offre de soin et de mieux financer les établissements dans notre pays depuis plusieurs années, le CHU de Pointe-à-Pitre et confronté à des difficultés financières qui entrave son bon fonctionnement vous-même aviez mis en place un plan ambitieux d'accompagnement dont l'objectif était d'améliorer la qualité et la sécurité, la prise en charge des patients, mais aujourd'hui, Madame la Ministre, la situation s'est aggravée suite à l'incendie qui a frappé l'établissement de Pointe-à-Pitre le 28 novembre dernier en effet, ce sinistre implique non seulement la remise en état des locaux mais également une stratégie pour préserver les effectifs, les effectifs des médecins soit dit en passant de 50 pourcent des urgentistes sont sur le point de quitter le CHU, cela s'ajoute aux difficultés classiques de recrutement de spécialistes et ne favorise pas la bonne prise en charge des patients, ce qui entraîne autour de fuite, important, de ce fait, le plan annoncé apparaît aujourd'hui insuffisant, il doit donc être adopté pour répondre à l'urgence de la situation, par ailleurs, il était pourtant pour garantir un niveau de trésorerie constante qui assurer la fluidité des approvisionnements, médicaments et autres fournitures de mensualiser le versement des aides cette action contribuerait au bon fonctionnement du CHU de Guadeloupe Maddalena Ministre vous connaissez mon engagement dans le domaine de la santé, ma préoccupation constante concernant l'amélioration de l'état de l'offre de soins de nos territoires, ma question est donc la suivante sans attendent l'application de la nouvelle réforme concernant le financement des hôpitaux et face à cette situation inédite : quelles mesures financières complémentaires comptez-vous mettre en oeuvre pour solidifier la trésorerie du CHU de Pointe-à-Pitre dépossédé aux réparations et acquisition d'équipements nécessaires. Pour vous répondent : la parole réclame Madame la ministre des solidarités, de la santé, vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Dominique Théophile, vous avez raison, l'accident qui a touché la Guadeloupe, le CHU cet incendie du 28 novembre a été dramatique, heureusement sans drame humain, il a énormément fragilisé l'offre de soin de la Guadeloupe, et vous savez, j'ai pris ce sujet à bras le corps, je me suis rendu sur place, 48 heures après, je tiens d'ailleurs à souligner l'extrême sang-froid des professionnels de ce CHU qui ont évacué que la quasi-totalité du CHU sans blessés à la présidente de la Seine Madame Suzie Duflot qui opéraient pendant que la fumée envahissait son bloc opératoire au directeur Monsieur Thépot qui met tout en oeuvre pour remettre en état ce CHU, nous avons fait livrer, vous le savez, un hôpital de campagne un hôpital militaire, mais il faut évidemment que les finances soient au rendez-vous et nous sommes là, nous y travaillons, j'ai décidé d'allouer au CHU de la Guadeloupe 69 millions d'aides exceptionnelles en 2017 soit 20 millions d'euros supplémentaires que le montant déjà perçu en 2016, qui était déjà à un niveau très exceptionnel. C'est 20 millions d'euros d'euros supplémentaires permettront d'acquérir sans délai les équipements et prestations de travaux nécessaires à la remise en état et notamment la achat le la location de bloc opératoire, par ailleurs, je suis en mesure de vous confirmer que tout comme en 2017 les aides en trésorerie continueront d'être mensualisé en 2018, enfin, je souhaite que les Guadeloupéens retrouve rapidement une offre de santé à la hauteur de leurs besoins et l'activité normale du CHU je souhaite que ce CHU soit remis en état, en attendant la livraison du nouvel hôpital en 2020, 2, vous savez que les marchés publics ont été lancés, il s'agit d'un investissement massif de l'État pour 580 580 millions d'euros, le nouveau CHU sera livré en 2020, vous pouvez compter sur mon entière détermination pour la santé des Guadeloupéens, je vous remercie. Merci, la parole est. à notre collègue Gisèle Jourda pour le groupe socialiste et républicain. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture j'associer mes collègues Henri Cabanel et Franck Mantaux, j'ai ainsi que les sénateurs issus de tous les bords qui vous emmène tefois sollicité sur le zonage des zones défavorisées, oui, nous vous avons alerté et relayer auprès de vous, de vos services les inquiétudes de nos agriculteurs qu'allait-il aujourd'hui car c'est bien aujourd'hui que vous arrêtez la carte définitive des nouvelles zones pour la transmettre à Bruxelles le 1er mars cela réduit le Tir, faut-il dire qu'il nous reste 14 jours pour vous convaincre, ou convaincre le président de la République, alors Monsieur le Ministre, éclairez notre lanterne car évoluer dans cette carte, quel est son périmètre quels critères avez-vous retenu, pouvez-vous nous le laisse poser vous dites avoir travaillé avec concertation équilibré clarté tellement de concertation, d'équilibre et de clarté que les agriculteurs touchés et les élus concernés ont manifesté manifestent encore sur nos routes, autoroutes et au coeur des départements aussi divers a de Gers Ariège ont Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées Tarn-et-Garonne le Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Loiret environ Val-de-Loire, Deux-Sèvres et j'en passe, avez-vous autour du compte de leurs revendications et de la réalité du site de ces situations sur ces territoires défavorisés chez moi, dans l'Aude, en Occitanie, les agriculteurs de la Piaget durable est-ce que le du zonage, alors que les électeurs et se sont vu refuser par les services de l'État, la transmission de l'étude de l'île et ces critères sélectifs 24 communes, 55 exploitations touchées est ce normal face à ces inquiétudes et angoisse croissante, dites-nous, Monsieur le Ministre, combien de communes en été dans le périmètre et comment vous comptez accompagner dans la durée,

activité. Ce ministre, vous avez la parole. Merci, merci, monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, Jourdain, vous avez raison, vous nous avez alertés mais peut-être auriez pu plutôt que de nous alerter, faire le travail parce que le zonage sur lequel nous travaillons madame la sénatrice à 40 ans parce que depuis 15 ans, la Cour européenne des comptes à demander à la France de revoir ce zonage et parce qu'au fond la couardise permet toujours de laisser à d'autres la responsabilité de mettre en oeuvre les injonctions c'est ce gouvernement qui, madame la sénatrice la met en oeuvre, mais Madame la sénatrice, je ne doute pas de votre volonté et de notre conscience que je partage sur celles et ceux qui, exploitant agricole sortiront du bénéfice des aides des FDS et de lycéens, chaîne, je suis un élu des Alpes-de-Haute-Provence et je sais l'importance dans la ruralité dans la montagne de laisser madame la sénatrice quand je regarde la carte de France telle qu'a été présenté à l'ensemble de la profession, je constate que 3555 communes Net vont rentrer dans le bénéfice du nouveau zonage quand je regarde votre département et j'ai apprécié la méthode de Jean-Michel Blanquer avait je vais la faire mienne quand je regarde département d'c'est un frisson aperçoit que aujourd'hui à peu près une centaine de communes sont bénéficiaires de ce classement, la demain, ce seront 100 de plus et je ne doute pas, Madame la sénatrice, que non seulement vous allez retourner voir les agriculteurs sur ce territoire pour dire que l'amélioration de la situation, vous la devez non pas votre intervention à l'instant présent, mais Stéphane Travert et peut-être même que le courage politique pourrait nous amener à aller les voir et leur dire : voilà pourquoi depuis des années, nous n'avons pas eu le courage de refaire sa cartographie et que, sans nouvelles communes en bénéficient aujourd'hui, dans votre département. Paroles et maintenant notre collègue Jérôme Bosch. Pour le groupe républicain. Monsieur le président, mais, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie. Le président de la République avait annoncé une réforme des retraites par points. Nous n'avons vu dès janvier que les point de CSG supplémentaire. Je cite le président toujours en mai dernier aux plus aisés, les retraités, je demanderai un effort. La retraite moyenne est 2376 euros soit 100 euros de moins que le SMIC, vous prenez directement 300 euros de plus chaque année dans les poches de 2 tiers des retraités est cela les plus aisés, ceux qui ont travaillé toute leur vie pour un salaire modeste, ceux qui ont connu des carrières incomplètes, liée au chômage de masse. Ce nouveau renoncement n'est hélas que l'illustration de vos raté technocratique en matière de pouvoir d'achat, la neutralité fiscale annoncée s'est muée en simple neutralité sur le paquet de cigarettes, mais toujours avec des taxes supplémentaires, elle s'est muée en hausse des carburants, d'aujourd'hui et de demain pour le banlieusard toujours obligé de prendre sa voiture pour aller travailler ou pour le provincial qui obligé de la prendre tout simplement pour vivre et je ne parle pas. Du nombre et du montant des amendes de stationnement qui explose. Toutes ces classes moyennes oubliée voire inconnue du gouvernement souffre d'un pouvoir d'achat fortement entamé en ce début d'année, menaçant la croissance enfin retrouvée à cette triste réalité humaine s'ajoutent les annonces de l'INSEE sur la baisse générale du pouvoir d'achat qu'un de vos collègues s'est permis de dénoncer toute honte bue, alors Monsieur le ministre ma question est simple pour corriger radicalement les erreurs qui découle du tropisme par trop technocratique et parisien du gouvernement, quelles mesures allez-vous prendre dès ce printemps pour un partage enfin juste des fruits de la croissance. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le flatteur, votre question est intéressante puisqu'elle porte sur la question du pouvoir d'achat et de la manière dont nos concitoyens peuvent vivre aujourd'hui est envisagé de construire leur avenir, vous avez cité la question de la CSG, la CSG a été augmenté, il est vrai, elle a été compensée pour l'ensemble des salariés du secteur privé, par une diminution de 3,15 des cotisations chômage et maladie, ce qui se traduit par une augmentation du pouvoir d'achat, pouvoir d'achat qui sera amplifiée avec la 2ème vague de baisse des cotisations au mois d'octobre et qui sera aussi amplifié dans la même période, avec la mise en aviez dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des ménages cette CSG a été augmentée pour les fonctionnaires, et nous avons veillé à ce que cette augmentation soit totalement neutralisé et neutraliser d'abord parce que nous avons prévu, pardonnez-moi une indemnité compensatoire, dont les modalités ont été fixées par un décret du 31 décembre elle a été prévue aussi parce que nous avons fait en sorte que les employeurs publics et les moyens de compenser cette augmentation de CSG par l'inscription de 290,5 millions d'euros de crédits dans le budget de l'État et par la diminution de la cotisation employeur maladie de 11 heures 59, 70 pourcent pour les autres employeurs et elle a été augmenté, il est vrai pour les retraités avec une particularité, c'est que cela s'applique uniquement à partir d'un revenu fiscal de référence supérieure à 14404 euros pour une personne seule, qui correspond à une pension mensuelle nette 2394 euros pour une personne seule depuis 65 ans, et 2289 euros pour une heure, une personne retraitée de moins de 65 ans, pour les 2 tiers des retraités, pour les 2 tiers des retraités, la mesure sera neutre, note parce que d'abord il y a exonération pour une partie d'entre eux, et par ailleurs, le montant moyen dégrèvement de la taxe d'habitation permettra de neutraliser cet aspect Monsieur le Sénateur, permettez-moi de vous dire que les fruits de la croissance sont partagés, partagés équitablement, ils le sont, ils continueront à l'être, et les Français le savent et ils savent que le projet présidentiel s'appliquera progressivement à leur Avantage, permettez-moi si tu vois conclure que ce que nous mettons là est bien différent de ce qui était prévu par d'autres, avec l'augmentation annoncée 2 points de la TVA, ce qui aurait correspondu si cela avait été mise en oeuvre par votre famille politique d'accroissement de la fiscalité de 13 milliards d'euros. La parole est maintenant notre collègue Martin décidera pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre monsieur le 1er ministre la misère existe dans notre pays des femmes et des hommes vivent dans la rue et depuis le début de l'année, plusieurs SDF sont morts à Paris : nous devons tous lutter contre cette réalité, c'est une question d'humanité lorsque j'entends monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État a déclaré que le nombre de personnes isolées, dormant dans la rue en Île-de-France correspond à une cinquantaine je m'indigne et je l'invite à aller à l'eau rencontrent dans une interview récente lui Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, révèle que les préfets excluerait de leur comptage des personnes sans abri, les célibataires et ceux qui vivent sous une tente, sans doute, les préfets se sentir lié par la promesse du président de la République, disant qu'il n'y aura plus personne dans la rue, à la fin de l'année 2017, nous sommes en 2018 et hélas cette promesse non plus n'est pas tenu, pensez-vous, Monsieur le 1er Ministre comme Julien Denormandie qu'il n'y a que 50 personnes qui dorment dans la rue en Île-de-France, pensez-vous, Monsieur le 1er ministre comme le député de votre majorité Sylvain Maillard que l'immense majorité de SDF passent la nuit dehors par choix, pensez-vous, Monsieur le 1er ministre que le président de la République, emporté par sa communication a tenu sa promesse, monsieur le 1er Ministre ne pensez-vous pas que nous sommes face à 3 5 News.

Je crois que, face à des situations qui sont, je l'ai dit tout à l'heure des situations de drame. De la misère, de la solitude, cette polémique sur les chiffres tout à fait déplorable, elle est déplorable, je ne me suis jamais engagé sur cette question de chiffres, je sais que nous partageons tous, ici et ailleurs au gouvernement à l'Assemblée nationale dans nos collectivités le même objectif, c'est moi, il y a eu le moins possible de nos concitoyens dans la rue le moins possible, sans abri, d'autres l'ont fait sous tous les gouvernements, et je dis que cette polémique, elle est déplorable, car quand vous dites que nous donnerions désordre à des préfets pour cacher la vérité, jamais nous ne ferons ça jamais, parce que je respecte, nous respecterons les préfets dans ce pays qu'ils font le maximum d'eau sommes chaque semaine avec le secrétaire d'État Julien de Normandie en conférence avec avec les 13, préfet de région, pas pour leur dire de changer les chiffres pour leur dire l'attention du gouvernement pour leur dire : la nécessité de faire en sorte qu'il n'y a plus l'enfant qu'il n'y a plus de famille dans la rue, effectivement, il y a eu des résultats positifs par rapport à ça, mais il y a encore beaucoup trop d'hommes et de femmes dans ce pays qui sont sans abri et encore dans la rue alors que l'on fasse de ce sujet et de phrases qui peuvent être échangés dans des maximales des sujets de polémique, je vous le dis en face c'est détestable. Madame de Chirac. De grâce, Monsieur le Ministre attelez-vous vraiment au vrai sujet au travail de fond et cessons de polémiquer là-dessus et, ensemble, ensemble, faisant mentir Bertold Brecht qui disait si les puissants de la Terre sont capables de provoquer la misère, ils sont incapables d'en supporter la vie, nous comptons sur vous tout de même. samedi, séance de questions d'actualité, auront lieu mardi, merci Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, la séance est suspendue, elle sera reprise à 16 pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, la séance est suspendue.

Sa collègue, la séance est reprise, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'orientation et la réussite des étudiants

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission mais, chers collègues, le vote des conclusions d'une CMP réussi est toujours un moment fort, émouvant, mais cet après-midi ne fait pas exception. Je voudrais tout d'abord à Mercier et le rapporteur de l'Assemblée nationale, il y pour son travail pour la correction de ces propos à mon encontre et puis pour la réussite de cette CMP, je voudrais aussi remercier Madame la ministre pour son écoute pour le respect de cette belle institution de ce toute de s'assembler d'autant plus que la réussite de ses thèmes de cette CMP était loin d'être une évidence au début de l'examen de ce projet de loi, je m'étais d'ailleurs engagé dès l'Automne auprès de mes collègues a être un rapporteur vigilant et je me suis astreint, c'est ainsi que l'essai n'a pu indiscutablement apposé sa marque de fabrique sur ce texte. En séance publique la semaine dernière, nous y avions rappelé les principes auxquels nous sommes attachés en matière d'enseignement supérieur, tout d'abord, primauté à l'insertion professionnelle, car il est criminel de laisser des jeunes s'engager sur des voies que l'on sait sans issue, c'est au nom de ce principe que votre commission avait proposé que les modifications des capacités d'accueil prennent en compte les Nasser sont professionnels observer de façon à éviter d'ouvrir toujours plus de place dans des formations, certes très demandés, mais sans débouchés professionnels, je sais, Madame la Ministre, que certaines syndicat se sont émus de cela

dans la loi, c'est chose parce qu'il faut aussi abandonner les prendre en compte, c'est une tout également au nom de ce principe que de nombreux amendements renforçant la prise en compte de la professionnelle des étudiants avait été adoptée par notre assemblée, à l'initiative de nos collègues, Guy et Max Brisson le 2ème principe qui a quitté notre travail, c'est le respect de l'autonomie des établissements, car nous devons faire confiance à nos établissements et à leur équipe dirigeante, ils sont bien souvent dans les dispositifs que les législateurs imagine les mieux placés pour évaluer et évaluer les situations il y apporter des solutions adaptées à la réalité du terrain, la loi LRU loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007 loi laquelle j'ai pu participer est une loi importante qui a marqué notre territoire en tout cas la l'université française et c'est au nom de ce principe que votre commission avait souhaité que l'établissement soit associé à la décision d'inscription dans une formation du candidat qui n'aurait eu aucune règle réponse positive à l'idée et à l'issue de Parcoursup, c'est aussi au nom de ce principe que nous avions proposé que les établissements puissent fixer librement les droits de scolarité des étudiants extra-communautaires, comme l'avait proposé notre collègue Olivier Paco le 3ème principe que nous avons souhaité défendent : c'est le principe de transparence car l'accès à l'information permet à nos jeunes de prendre des décisions éclairées pour leur avenir, c'est au nom de ce principe que la Commission avait proposé la publication des algorithmes locaux qui seront utilisés par les établissements pour classer les candidatures. C'est au nom également de ce principe que nous avons renforcé les obligations statistique des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi des établissements scolaires, comme le souhaitait notre collègue Stéphane Piednoir alors oui, mes chers collègues, je dois le reconnaître le texte que nous avons voté en CMP et que le gouvernement ne se mais ce soir, et en de nombreux points, bien différent de celui que nous avions voté il y a une semaine, plusieurs des apports du ciel parmi ceux que je viens de citer non plus n'ont pas passé le cap de la CMP, mais c'est la loi du genre, cela ne veut rien dire, que nous aurons donc renoncer à nos convictions que nous aurions accepté de signer un blanc-seing au gouvernement, nous avons décidé en conscience d'aboutir à un texte de comprimés de compromis avec l'Assemblée nationale, car il aurait été irresponsable de prendre en otage les quelque 850000 candidats qui ont déjà commencé à renseigner Parcoursup bien entendu, nous avons regretté l'étroitesse de ses calendrier parlementaire dans lequel nous avons été en Syrie, mais notre sens de l'intérêt général, monsieur Assouline nous a naturellement conduit accepter le caractère d'urgence de cette réforme et les contraintes qui en découlent et vous avez l'obligeance de le rappeler, la semaine dernière à cette même tribune, Madame la Ministre, sur de nombreux sujets, le Sénat a été précurseur et je vous en remercie, du régime du régime de Sécurité sociale des étudiants. CAC grâce à Catherine Procaccia sur l'orientation vers et dans le supérieur grâce à Guy Dominique Kennel sur la sélection à l'entrée dans le second cycle grâce à Jean-Léonce Dupont permettez-moi de penser, et même d'espérer que le Sénat aura été cette fois encore, précurseur dans ses travaux et que de nombreux sujets que nous avons soulevés dans ce timide dans cet hémicycle et qui n'ont pas trouvé grâce aux yeux de nos collègues députés progresseront dans les mois à venir, je vous en remercie. remercie. Cher collègue, la parole est maintenant mais. La Ministre Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation, vous savez la parole Madame 1 minuit. Madame Madame la présidente, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication Chère Catherine Morin-Desailly, monsieur le président

au coeur du projet de loi Orientation et réussite des étudiants, il y a une ambition, celle d'accompagner plus de lycéens et d'étudiants vers l'enseignement supérieur et vers la réussite, c'est l'épine dorsale de ce texte, c'est la boussole que je me suis fixé et c'est cette conviction que j'ai souhaité partager avec vous tout au long de l'examen de ce texte. Chacun le voit bien la massification s'est faite à l'école comme à l'université mais la démocratisation reste à faire l'accomplir et la réussir, c'est là le défi qui s'offre à nous, et c'est la raison pour laquelle au-delà des dysfonctionnements inacceptables qu'a connu la procédure d'entrer dans l'enseignement supérieur, le gouvernement a souhaité construire un plan étudiant qui saisissent dans sa globalité, la question de l'accès aux études supérieures, dans ses composantes pédagogique mais aussi le le plan étudiant c'est un bloc à bloc qui apporte des réponses concrètes à des questions concrètes qui ne sépare pas l'accompagnement pédagogique, les politiques de prévention et d'action en faveur de l'âge étudiant. Tout au long de la préparation et de l'examen de ce projet de loi, je me suis attaché à faire vivre le dialogue le plus large avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et des forces politiques représentées dans cet hémicycle, parce que je sais que l'enjeu est trop important et que l'avenir de notre jeunesse fait partie de ces grandes causes qui peuvent nous rassembler très largement. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité asseoir ce projet sur une base saine et solide en ouvrant dès le mois de juillet, une large concertation et en la conduisant tout au long de l'été. Ce dialogue gelé noué dès le 1er jour de ma prise de fonction, et je le poursuis jour après jour, parce qu'il est essentiel de continuer à partager chaque fois que nécessaire les points de vue et les attentes d'entendre les interrogations et de dissiper les incompréhensions, je sais que vous partagez cette conviction et sénatrices et messieurs les sénateurs et nos débats en ont témoigné, ils ont permis à chacun d'exprimer, dans le respect, ses convictions propres et d'entendre ce que l'ensemble des forces politiques avaient à dire, ce débat est légitime, il est nécessaire, il est sain dans une démocratie et c'est le rôle constitutionnel du Sénat que d'apporter ainsi un autre regard sur les orientations politiques du gouvernement. Lors de l'examen du texte en première lecture le Sénat a fait entendre sa voix, nous avons eu parfois des divergences, chacun a pu le constater, mais nous avons aussi l'accord collectivement d'avancer et je tenais à vous en remercier, mesdames et messieurs les sénateurs. Nous sommes maintenant arrivés au stade de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire et je me réjouis que très sincèrement que celle-ci était conclusive et je tiens à en remercier la présidente de la commission Catherine Morin-Desailly, le rapporteur Jacques Grosperrin et l'ensemble des membres de la CMP dans les 2 assemblées, d'avoir su travailler dans un ex-dans un esprit constructif. Car, quelles que puissent être nos divergences, ce qui nous rassemble, c'est le souci de tourner la page du tirage au sort, et de mieux accompagner les futurs étudiants vers l'enseignement supérieur et vers la réussite, et comme je les rappeler lors de la présentation du texte sur de nombreux sujets, l'orientation, le tirage au sort, mais également le régime de sécurité sociale étudiant, le Sénat a été précurseur sur de nombreux points nous sommes ainsi parvenu à améliorer ensemble le texte présenté par le gouvernement, qu'il s'agisse du fait d'accueillir sur Parcoursup toutes les formations dès 2019, de renforcer les informations mises à disposition des futurs étudiants sur la plateforme d'élargir aux étudiants âgés de 25 à 28 ans, les actions de prévention mis en place dans le cadre de la réforme. Le rôle de vos commissions et de vous rapportera a été décisif et je tiens à le saluer comme je salue et remercie l'ensemble des sénateurs issus des différents groupes politiques qui ont tous contribué à enrichir et améliorer ce texte, nous avons eu aussi des désaccords relève 3 principaux. Le 1er tenait à la signification de l'autonomie des universités, nul n'est plus attaché que moi, vous le savez, et je suis convaincu que les universités sont fortes, lorsqu'elles sont autonomes et qu'elles ont les moyens de construire et d'affirmer un projet à la fois pédagogique et scientifique. Mais la régulation apportée par l'État doit être à la hauteur de cette autonomie afin de garantir le respect des attentes collectives qui sont les nôtres et le respect de principes fondamentaux, ce n'est pas une posture théorique, c'est une conviction pragmatique car c'est bien l'État, par exemple, qui est le garant de l'ouverture de l'enseignement supérieur à l'ensemble des étudiants, et c'est pourquoi dans la procédure Parcoursup c'est le recteur qui doit pouvoir inscrire les futurs bacheliers lorsqu'ils n'ont pas de propositions. Vous avez souhaité la commission mixte paritaire a rejoint sur ce point, le Sénat, que cette inscription d'Office puisse être précédée d'un dialogue et, bien sûr, je suis favorable, comme je suis favorable à l'idée, issu des travaux de la CMP de permettre aux établissements de nourrir ce dialogue en faisant à leur tour des propositions. Ce dialogue est nécessaire comme il est nécessaire que le recteur puisse in fine et prononcé l'inscription et je salue donc la rédaction issue des travaux de la CMP, qui me paraît parfaitement équilibré. 2ème point de divergence, les critères de fixation des capacités d'accueil, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours, vous aviez souhaité, à l'initiative de votre rapporteur corréler directement cette décision au taux de réussite et d'insertion professionnelle j'ai eu l'occasion de le dire, le gouvernement entend le souci exprimé par le Sénat de donner toute sa place à la mission d'insertion professionnelle reconnue depuis 2007, qui est l'une des 4 missions de l'université, à côté de créer de la connaissance, la diffuser et diffuser la culture scientifique et technologique de nombreux amendements déposés en ce sens ont permis de consolider les dispositifs existants et figure dans le projet de loi issu de la CMP pour autant une corrélation directe entre ses capacités d'accueil et les taux de réussite et d'insertion, c'était prendre le risque d'installer une forme d'. L'équation Nice Nisman alors même que nous voyons tous les jours qu'émergent de nouveaux métiers, de nouveaux besoins de qualification par exemple dans le domaine du numérique, je sais que ce sujet vous est cher. Nous avons beaucoup échangé à ce sujet avec le rapporteur Jacques Grosperrin, je veux le remercier de la qualité de ce dialogue sur ce point comme sur tous les autres. a aussi la CMP a permis de clarifier les choses, en mettant en avant la notion de perspectives d'insertion professionnelle, mais en prenant en compte aussi le projet de formation et de recherche des établissements et les attentes des étudiants. Cette rédaction, me paraît plus équilibrée et permet de prendre en compte l'intégralité des attentes exprimées, celle des étudiants aussi car, vous le voyez, chaque jour, dans vos territoires le choc démographique et là et nous avons le devoir d'y répondre en accompagnant, guidant les futurs étudiants bien sûr mais aussi en ouvrant largement les portes de notre enseignement supérieur, y compris celui qui est plus professionnelle ou plus professionnalisant à l'ensemble des étudiants. C'est la marque du Sénat que de pouvoir exprimer ses différences de points de vue tout en faisant oeuvre législative utile et qu'elle est bien le cas, et le texte de la commission mixte paritaire, tout comme vos travaux sont là pour en témoigner. Vous avez l'âme de messieurs les sénateurs, saisi tout l'enjeu de cette réforme et je tenais à vous en remercier car l'important, c'est bien de répondre aux attentes des futurs étudiants et de leurs familles qui ont besoin de clarté, de sérénité pour faire leur choix en toute responsabilité. Si vous suivez les conclusions de la CMP votre vote nous permettra de clore le chapitre de la refondation juridique de l'accès à l'enseignement supérieur pour ouvrir celui de la mise en oeuvre de la campagne d'affectation 2018, je sais que les attentes et les exigences qui pèse sur le gouvernement sont fortes. Sachez que je suis déterminé à et répondre avec énergie, calme, sérénité, dans l'intérêt de notre jeunesse, je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Colette Mulhouse pour les indépendants.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la Commission, monsieur le rapporteur, mais chers collègues. L'Assemblée nationale et le sénat ont trouvé un compromis mardi dernier autour d'un nouveau texte relatif au projet de loi Orientation et réussite des étudiants. Il convient tout tout d'abord de saluer le travail des rapporteurs Gabriel Attal et Jacques Roux Perrin qui nous conduit aujourd'hui à examiner un texte équilibré, respectueux des avis et des des uns et des autres et surtout les c'est essentiel à la refonte de l'enseignement supérieur en France, c'est l'occasion de redire en quelques mots l'état inadaptée de notre système d'enseignement supérieur et de l'urgence à le réformer un manque criant de diplômés en sciences, technologie ingénierie et mathématiques des débouchés très variables d'une formation à l'autre, un choix dans l'accès à l'enseignement supérieur, beaucoup plus large, mais en conséquence des parcours parfois moins cohérent et enfin une filière professionnelle très peu suivie, avec seulement 23 pourcent des 15 19 ans, soit une proportion de 6 points inférieurs à lui 22. Face à tous à cette situation, députés et sénateurs ont agi avec raison en trouvant un accord entre les textes de nos 2 assemblées suivant l'esprit de responsabilité évoquée par le rapporteur, la CMP a donc abouti à un accord qui empêchera que la nouvelle plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur Parcoursup ne soit bloqué par un retard dans le la l'adoption de ce projet de loi, je crois que nous pouvons nous en féliciter. Plusieurs points restent en débat et nous opposer à nos collègues de l'Assemblée nationale : premièrement, la problématique des bourses et des dispositifs de délivrance chiffré à hauteur de 2 milliards d'euros par an pour l'État, ces bourses sur critères sociaux ne peuvent être délivrés sans vérification, la CMP, propose de mettre en place une obligation d'assiduité pour les étudiants boursiers, c'est une première étape dans leur responsabilisation. Deuxièmement, la question de l'insertion professionnelle que mon collègue de groupes Daniel Chassain, évoquée hier encore lors des débats sur le projet de loi de ratification des ordonnances relatives au dialogue social, inutile d'envoyer nos étudiants dans les filières sans débouchés professionnels, la CMP trouve là encore un compromis raisonnable, l'ouverture de places sera conditionnée par les perspectives d'insertion professionnelle et l'évolution des projets de formation de l'établissement, troisièmement, les droits d'inscription des étudiants étrangers, notre groupe avait posé sur la table une proposition d'amendement autorisant les universités à majorer les droits d'inscription d'étudiants étrangers hors Union européenne, la CMP n'a malheureusement pas retenu cette proposition mais nous pensons utile de la retenir et de la proposer à nouveau à l'occasion des débats financiers de l'année 2018 puisque la question de l'autonomie fiscale des établissements de bain d'enseignement supérieur. Sera très rapidement quatrièmement et dernièrement, la question du droit de véto de l'établissement. Le projet de loi mettait en place une procédure dite du dernier mot au du au candidat, obligeant le recteur à faire une proposition de formation aux candidats sans inscription à l'issue du parcours normal ce principe n'était pas tenable et l'est obligé nous rectorat à traiter des milliers de dossiers au coeur de l'été, la CMP met en place une formule intermédiaire obligation du rectorat de respecter les capacités d'accueil et obligation pour le candidat d'accepter pour le candidat d'accepter un parcours personnalisé si l'établissement le juge nécessaire. Madame la présidente, Madame la Ministre, mais, chers collègues, ce projet de loi ambitieux est une étape essentielle du projet de rénovation de l'école républicaine et de la formation dans notre pays, conduits par le président de la République par le ministre de l'Éducation nationale et par la ministre de l'enseignement supérieur, l'étape que nous franchissons aujourd'hui, nous la faisons pour les générations futures pour nos enfants, nos petits-enfants et une arrière-petits-enfants en leur donnant la possibilité de réussir dans le monde de demain en réformant les procédures d'accès à l'enseignement supérieur et en simplifiant le régime de sécurité sociale étudiant ce projet de loi offre : lisibilité efficacité et fonctionnalités un système à bout de souffle permettons lui de prendre un nouveau départ afin d'assurer la reconstruction durable de notre pays et la relance de notre économie, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, les mutations de la société doivent être prises en considération par les décideurs politiques pour permettre l'accès de tous nos concitoyens, connaissance et au savoir des transformations structurelles liées à l'automatisation des tâches et au développement de l'Intelligence artificielle affecte parallèlement le marché du travail et l'emploi en profondeur, s'engager dans la voie du changement pour construire une société où les jeunes s'épanouissent et dispose des outils nécessaires pour s'adapter à ces bouleversements et d'un long travail qui reste à accomplir, l'université, un rôle central à jouer en la matière, pourtant comme exprimaient justement Jacques Chaban-Delmas en 1969 devant l'Assemblée nationale, nous ne parvenons pas à accomplir des réformes autrement qu'France semblant de faire des révolutions si le groupe RDSE s'est prononcé contre l'instauration d'une sélection aveugle à l'entrée de l'université, c'est parce qu'il a jugé qu'elle serait socialement discriminatoire et aggraverait les inégalités scolaires déjà très prononcées dans notre pays, notre groupe a donc tenté par ces amendements d'en atténuer les effets lors de l'examen du présent projet de loi à l'issue de la réunion, c'est de la CMP quelques avancées peuvent toutefois être salué la grande majorité des éléments qui présentait l'enseignement supérieur dans une logique essentiellement économique a été extirpé du texte c'est positif car le parcours d'orientation doit être capable à tout moment en fonction des aspirations de l'étudiant des capacités qu'il peut développer parfois tardivement ou encore de sa motivation pour ces raisons, nous estimons que l'orientation ne doit pas être élaborée exclusivement à l'aune des attentes présupposé des entreprises en première lecture, nous étions en particulier opposé à une détermination des capacités d'accueil directement corrélée au taux de réussite et d'insertion professionnelle des formations désormais la rédaction retenue par la CMP est devenue plus vague avec une référence aux perspectives d'insertion professionnelle au projet de formation et de recherche de l'établissement ou encore à l'évolution des projets de formation des candidats, ce dernier critère correspond mieux à ce que le RDSE à défendu, même si nous reconnaissons la faible portée législative de ces dispositions. Je me réjouis principalement que dans le cas de la dernière partie de la procédure de pré-inscription pour les candidats sans affectation, mais aussi dans la procédure devrait examens pour circonstances exceptionnelles, la CMP et tranché en faveur d'une décision prise par le recteur, respectant le principe de l'accès de tous les bacheliers au 1er cycle de l'enseignement supérieur, droit, un droit qui ne doit pas leur être retirée le Baccalauréat étant le 1er grade de l'enseignement supérieur, je salue également le maintien de notre amendement qui prenait en compte le projet de formation du candidat sans affectation, enfin, préserver l'objectif de maîtrise de la langue française et bienvenue, même si nous aurions préféré une concrétisation de ces dispositions purement déclaratoire dans le projet de modules d'accompagnement proposées par les universités je regrette en revanche la persistance de problèmes qui n'ont pas obtenu de solutions acceptables telles que le frein à la mobilité, l'accès aux universités parisiennes que constitue le pourcentage maximal de bacheliers hors académie, en particulier pour les bacheliers outre-mer, le sort des bacheliers professionnels et technologiques n'est pas non plus réglée et pourtant l'objet de cette loi porte également sur la réussite de tous les étudiants, l'amendement que nous proposions visant à établir un pourcentage plancher de ces bacheliers dans les filières STS et IUT a été rejeté par le Sénat, alors qu'il permettait d'apporter une première réponse, si l'on ne peut nier les améliorations apportées par le projet de loi par rapport à la situation actuelle, on se rend compte au fil des discussions que la très grande partie des candidats fera encore l'objet d'un traitement déshumanisée de la procédure par l'intervention d'algorithmes locaux, seuls ceux qui n'auront pas été les mieux classés bénéfique si d'une intervention humaine et la prise en compte du parcours extra-scolaires du bachelier instaure, j'insiste, des critères socialement discriminant et surtout dans un contexte de réforme du Baccalauréat, on ne voit plus très bien où l'on va avec la disparition des filières S L, ES, la mise en place d'un tronc commun de spécialités, le gouvernement s'engagera-t-il à revoir les critères de Parcoursup les universités ont subi dans un passé très récent, un sous-investissement chronique et des prélèvements par l'État sur leur fonds de roulement dans ce contexte, leur manque de moyens accroît non seulement le caractère sélectif de l'entrée dans les formations en tension mais impact aussi l'ensemble des étudiants lors dans leurs conditions de travail lors de l'examen de la loi relative à la sélection en master à l'université notre rapporteur avait souligné qu'il existe, je cite, un risque d'instituer une université à 2 vitesses entre des master de 1er choix sélectif et des master poubelle qui accueilleront des étudiants recalés, c'est exactement ce que nous craignons dès l'entrée en première année entre les filières en tension et les autres, avec ce texte pourtant la rentrée devrait se passer dans de meilleures conditions que l'année dernière et nous le savons, il s'agit de régler en urgence l'affectation des bacheliers dès la rentrée prochaine, le présent projet de loi que la grande majorité du groupe RDSE soutiendra aura au moins le mérite de parvenir à cette fin, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Antoine Karam pour le groupe, la République en. Madame

Madame la présidente. Madame la ministre, madame la présidente de la Commission, monsieur le rapporteur monsieur recoller avec ce projet de loi dont l'examen s'achève, nous allons répondre et vous l'avez dit, ici à l'attente insoutenable de 800000 jeunes qui préparent actuellement leur entrée dans l'enseignement supérieur, nous l'avons dit le contexte était unique et je crois néanmoins que nous avons su dans une forme d'urgence, il faut bien le reconnaître, rapporté des restes avec responsabilité, une réponse juste et efficace, nous avons tous reconnu ici l'injustice induite, aussi bien par le dispositif APB que par cette honte sélection par l'échec qui prévaut malheureusement dans nos universités. Nous avons tous mesuré l'urgence de cette situation devenue insupportable dont nous portons collectivement la responsabilité, à partir de ce constat partagé, je crois que nous avons su engager un travail de fond dans un esprit irresponsable nous débat était riche et ont parfois révélait des désaccords profonds je crois néanmoins qu'en dépit des les contraintes du chemin a été parcouru et cela dans le bon sens, ce texte marque bien l'importance de la navette parlementaire et du Sénat, nos discussions en commission mixte paritaire ont rapidement pris le chemin d'un accord et à ce titre, je salue la volonté du gouvernement la sagesse du Parlement tout particulièrement celle du Sénat, le travail accompli par notre rapporteur, cet incident que l'on arrive telle résultat dont il faut ne pas négliger l'importance cet accord préserve, je le crois, l'esprit du plan étudiant en assurant à chaque jeune une voix personnalisé vers la Russie, tout en préservant les apports du Sénat, affirmation de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et plus grande prise en compte de l'insertion professionnelle dans l'orientation des étudiants. Nous apportons non seulement une réponse à un flou menaçant mais nous offrons un meilleur accompagnement vers leur réussite à tous les jeunes dans leur diversité, cela étant dit, et par delà nos débats j'ai pour ma part la conviction que ce travail s'approfondira encore plus dans les mois, venir, il faut être conscient par conçue comme d'autres dispositions de ce texte prendront leur pleine mesure car l'épreuve du terrain au contact de l'humain, je pense d'abord à l'orientation, la plateforme Parcoursup ne réglera pas à elle seule, cette question et nous le savons bien nous discussions montrer qu'il s'agit là d'un sujet complexe qui nécessite un changement de paradis dès l'entrée au lycée, ce texte pourtant le mérite d'en poser les fondations du temps et de la pédagogie seront toutefois nécessaires en pratique pour aider chaque étudiant a façonné son projet je pense ensuite à l'affectation des derniers étudiants, nous avons trouvé ici un point d'équilibre satisfaisant en supprimant ce droit de véto du chef d'établissement profit d'une obligation pour le recteur de respecter les capacités d'accueil satisfaisant car il ouvre la voie à une plus grande fluidité et un dialogue que nous espérons, intelligent, il était donc impératif d'éviter tout risque de blocage au milieu de l'été, je pense aussi à la détermination des capacités d'accueil en prenant en considération les souhaits des étudiants, le projet des établissements et l'insertion professionnelle nous atterrissons à mon sens, sur un principe équilibrée des inquiétudes, elles ont déjà été exprimée depuis notre réunion de commissions, mais il faut le dire, l'enseignement supérieur n'est pas ici dévoyé, il en fait précisément ligne avec les objectifs fixés par l'article L 612,2 du code de l'éducation et à savoir je cite accompagné tout étudiant dans l'identification et la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et d'une spécialisation progressive des études dans un but professionnel s'il fallait, j'en conviens, se départir d'une vision trop adéquation ministre il y a un important de prenant compte tous les facteurs pertinents, là encore le terrain nous dira si nous sommes dans le vrai, mais je crois que nous devons faire confiance au recteur et à son rôle régulateur, je rappelle que le recteur et ne l'oublions jamais chancelier des universités, autre sujet retenu en commission mixte paritaire l'assiduité des étudiants, notamment des bourgs, si nous parvenons à une solution mesurée qui rappelle finalement ce qui existe déjà, permettez-moi toutefois d'exprimer mon désaccord avec l'idée selon laquelle les étudiants boursiers seraient moins assidues que les autres pour dire vrai, et parler encore une fois d'une expérience de terrain, j'ai même la conviction que l'absentéisme touche tous les étudiants, et plus particulièrement ceux qui ont été mal orientées, qu'ils soient boursiers ou pas,

je pense enfin à la contribution unique cela la pratique nous dira si elle permet une amélioration concrète une diversification des actions de vie étudiante, j'ai évoqué le cas des étudiants ultramarins, j'espère que, d'une attention par spécifique et la collègue la lundi sera rapporter à leur accueil avec des actions dédié au sein de chaque établissement, il est certain que l'examen de ce texte a suscité une forme de frustration quand nous amener vers d'autres questions, je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait de ce plan étudiant une réforme aussi passionnante qu'exigeante dans un autre exercice, nous serons appelés à réfléchir sur l'apprentissage je formule le voeu que ce travail de ce travail plutôt sortira une solution ambitieuse et complémentaire à celle que nous votons aujourd'hui dans les messieurs, mes chers collègues, vous l'aurez compris les élus du groupe de la République en marche, nous voterons le présent texte avec de grands espoirs pour notre jeunesse, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, au sortir de la commission mixte paritaire, le sentiment qui prédomine, celui de la déception. Déception car ce projet de loi avait pour finalité de favoriser l'orientation et la réussite des étudiants, comme le souligne son attitude malheureusement l'intérêt des étudiants a été progressivement perdu de vue au cours des discussions au profit d'autres considérations désormais n'est plus l'objectif principal est fondamentale de ce texte, premièrement, d'orientation, il n'en a finalement été faiblement question au final, je n'ai pas reprend les développements que j'avais formulée lors de la discussion générale sur le texte, mais il est regrettable et même frustrant, j'ai entendu parler de frustration de ne pas avoir pu mener une réflexion beaucoup plus approfondie sur le sujet cloisonner ainsi notre réflexion empêche de penser globalement une politique de l'orientation ambitieuse qui créerait un continuum y entrent le secondaire et le supérieur, or ce manque de liant et précisément un des facteurs responsables de l'échec des étudiants en licence, le projet de Loire et puis aborder cette problématique, il aurait pu dessiner des pistes, il n'en a rien été, on était bien sûr un texte d'affectation et non d'orientation. Le bon sens commande pourtant de rappeler que la plupart des lycéens font des choix presque quasiment à l'aveugle, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais approché les matières qu'ils vont étudier dans le supérieur, au mieux, ils en ont une idée savante textuelle mais aucunement sensible, même si en terminale sont amenés à réfléchir davantage à leur orientation et c'est une évolution évidemment positif qui est en train de se passer, mais rien d'remplacera la mise en situation, lors de la 1ère année de licence car c'est celle-ci qui valide ou même invalide le projet d'orientation, par conséquent, il y a bien un continuum évident entre l'année de la terminale et la première année dans le supérieur, où le projet imaginé se confrontent en fait à la réalité des faits, c'est pour ça que ce continuum aurait dû être l'axe majeur d'une politique d'orientation en faveur de la réussite des étudiants il appliquait de changer radicalement de regard sur la première année à l'université en imaginant peut-être en commun passerelle en somme en permettant à l'étudiant peaufiner de parachever son projet d'orientation, nous aurions c'est vrai, mais ouvrir le débat, c'était le sens de certains de nos amendements, il n'en a rien été en introduction, j'évoquais notre déception à l'égard du texte issu de la CMP, en effet, lorsque le projet de loi est arrivé en débat au Sénat, nous ne l'avons bien sûr aucunement rejeter en bloc ce que nous souhaitions, c'est que les conditions soient réunies pour assurer la réussite de tous les étudiants, et c'est pour cette raison que nous avons soumis plus d'une trentaine d'amendements afin d'améliorer afin de valoriser les dispositifs d'accompagnement mis en oeuvre par les établissements afin d'améliorer la procédure dite de dernier recours pour les candidats qui n'avaient aucune affectation la majorité sénatoriale, on le sait, a fait évoluer le texte dans une direction complètement contraire à nos attentes, ce qui surprendra assez peu mais aussi antinomique à la volonté, je pense, initialement exprimée par le gouvernement, sur certains points du projet de loi, j'y reviendrai, il s'ensuit que nous ne pouvions pas, nous ne pouvions que qui se trouvait totalement dénaturé par les modifications apportées par la majorité sénatoriale, nous n'étions plus dans le jeu, une logique de réussite de l'ensemble des étudiants, mais bien dans une logique de sélection revendu assumer ce ne sont plus les étudiants qui choisissaient leurs sur université et qui bénéficie, éventuellement des dispositifs d'accompagnement, c'était les universités qui finissait pas recruter les étudiants de leur choix, une telle logique comme je l'ai exprimé en première lecture, c'était clairement entaché la promesse républicaine, alors oui nous attendions que la CMP quel rééquilibre le texte et nous sommes d'autant plus déçu que ce rééquilibrage n'a eu lieu qu'à la marge pour étayer mon propos, je prendrai 2 exemples concrets qui constitue, pour notre groupe politique des lignes en en 1er lieu : il s'agit de la manière de déterminer chaque année, les capacités d'accueil des formations du 1er cycle initialement, rappelez-vous, mais chers collègues était inscrit un principe général dans le projet de loi du gouvernement selon lesquelles ses capacités était, je cite, arrêtés par l'autorité académique après proposition de chaque établissement, nous y étions favorables, la majorité sénatoriale a souhaité préciser que ces capacités tiennent compte des taux de réussite et d'insertion professionnelle observer pour chacune des formations alors que notre système devrait faire preuve d'une souplesse manifeste pour adapter ses formations, eu égard à la rapidité des mutations qui traversent nos sociétés par l'intermédiaire du numérique, mais pas seulement l'Intelligence artificielle, le risque était bien de figer les offres de formation de scléroser la dynamique académique, voire même d'empêcher tendanciellement, les étudiants d'intégrer des filières d'avenir, ce qu'on a appelé beaucoup dans nos débats, les métiers de demain, in fine, hé bien que compléter la rédaction de compromis issu de la CMP, ces fameuses je ne comprends toujours pas perspectives d'insertion professionnelle des formations à à l'aune de la mesure des capacités d'accueil demeure un peu alambiquée incertaine d'un point de vue juridique et je l'ai déjà entendu et finalement, elle ne change rien sur le fond car on y retrouve l'adéquation entre l'offre et les besoins qui est contraire à l'objectif même de l'université et cette formulation aux incidences si notable est le fruit d'un compromis entre la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale est vraiment éloigné du texte initial, nous ne pouvons l'approuver la seconde illustration sur laquelle je désire prendre appui a trait à la procédure dite de dernier recours qui a pour but d'inscrire dans une formation, vous le savez, un étudiant qui n'aurait aucune affectation à l'issue de la saisine initiale de ces la la rédaction originale ne semblait pas optimales, mais l'article rédigé maintenant est pour nous inacceptable, nous avons toujours insisté sur le fait que l'équilibre de la réforme proposée par le gouvernement reposait en grande partie sur le recteur qui en est le garant, certes la CMP est revenu à cette idée, en conférant de nouveaux recteurs c'est vrai le rôle essentiel d'affecter un candidat dans une formation tout en supprimant le droit de véto les l'établissement dans cette procédure, c'est une bonne chose mais mais il y a un mais la rédaction Nouvelles de cet article et je l'ai encore relu n'accorde pas la confiance et la souplesse nécessaire aux recteurs dans le cadre du dialogue avec les du dire afin de lui trouver une formation qui corresponde à ses souhaits et de plus c'est ajouter l'obligation de oui ici qui durcit encore davantage la procédure de dernière chance chance s'ainsi qu'on a sur le droit à chaque étudiant poursuit ses études supérieures, est-ce ainsi qu'on fait primer l'intérêt de l'étudiant sur la régulation des flux l'opérationnalité d'un système où le manque de places dans les établissements est ainsi qu'on recherche réellement la réussite de tous les étudiants, je ne le crois pas, ainsi, bien qu'était retiré l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, nous ne pouvons souscrire au projet de loi issu de la CMP l'adage veut que la précipitation soit mauvaise conseillère, sûrement Madame la Ministre, était-il nécessaire pour vous d'obtenir un accord rapide entre les 2 chambres afin de donner une base légale à Parcoursup qui est d'ores et déjà rentrer en vigueur, sûrement, il y avait-il urgence mais cette urgence de se régler au détriment de l'intérêt des étudiants non seulement je le crois pas, mais je le regrette sincèrement que nous sur votre projet de loi que nous sommes amenés à nous prononcer ce soir, c'est sur un compromis excessivement bancal à forte insécurité juridique et empreint d'une tonalité et d'un esprit qui ressemblent finalement étrangement à ceux de la majorité sénatoriale et qui ne nous conviennent pas, en conséquence, nous voterons contre le projet de loi issu de la CMP, qui n'est décidément plus en faveur de l'orientation et de la réussite des étudiants, c'est un vrai rendez-vous manqué, merci.

la présidente, Madame la Ministre. Mesdames et messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire réunie pour examiner le projet de loi relatif à l'orientation et la réussite des étudiants est parvenu à un accord équilibré qui préserve les apports du Sénat est garanti garantira nous souhaitons un meilleur accompagnement des étudiants ainsi qu'une rentrée universitaire sereine cette année c'est un n', esprit de responsabilité qui a animé les parlementaires de la commission mixte paritaire, c'est ce même esprit qui nous a animés également lors des débats dans l'hémicycle, nous ne pouvions en effet rester laisser plus longtemps dans le flou et l'incertitude, tous les jeunes et leurs familles qui prépare à l'heure où nous parlons, leur entrée dans l'enseignement dans leur notre présidente de commission Catherine Morin-Desailly, ainsi que Jacques Grosperrin, rapporteur sur ce texte que je tiens à saluer pour leur travail et la qualité de nos échanges, l'ont rappelé cet accord préserve les grands apports du Sénat réaffirmation de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et plus grande prise en compte de l'insertion professionnelle dans l'orientation des étudiants. Le groupe Union centriste a voulu contribuer de manière responsable et intelligente au débat en apportant des améliorations au texte présenté par le gouvernement, je voudrais en retenir 3 cet après-midi, la première institut un comité éthique et scientifique auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour veiller au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de pré-inscription dans le supérieur, en effet, nous devons être attentifs à l'évolution et à l'utilisation dans le temps de la plateforme ainsi que des algorithmes locaux pour ne pas reproduire des dérives constatées avec APP la 2ème concerne la première année commune aux études de santé trop souvent réduite à une année de bachotage peu enrichissante pour les étudiants qui se heurte à ce couperet et ont le sentiment d'avoir perdu une année quand ce n'est pas 2, désormais, les étudiants pourront mener leur étude dans la filière qu'ils auront choisi tout le long de la licence, y compris en cas d'échec au concours de premières années des formations médicales, la 3ème en matière démographique, l'état se trouve placé devant une exigence qui relève parfois du défi : donner à tous les élèves sortant du lycée, une chance d'accéder à l'enseignement supérieur, le problème se pose d'une manière évidente à partir du moment où le nombre total de places disponibles est inférieur au nombre total de lycéens candidats à l'université, la pression démographique rend évidemment la situation critique et nous savons que c'est notamment sur ce point que les pouvoirs publics ont échoué ces dernières années, c'est pourquoi nous avons proposé que soit constitué un bilan annuel comportant un volet prospectif pour anticiper les évolutions démographiques, ces prévisions permettront d'évaluer l'adéquation entre le nombre d'étudiants attendus et les places disponibles dans les filières universitaires, elles éclaireront aussi le débat lors du projet de loi de finances, si les grandes orientations du texte vont dans le bon sens, il nous paraît insuffisant néanmoins sur plusieurs aspects et penser que la réforme de l'enseignement supérieur et celle de l'orientation, sur sa retraite à ce texte serait pour nous une erreur, le projet de loi ouvre des portes qu'il conviendra d'approfondir, à travers d'autres textes législatifs, c'est notamment la c'est notamment le cas de la question centrale, à nos yeux de l'orientation et aussi celle, tout aussi importante de l'organisation du 1er cycle de l'université, la licence encore très marquée par des schémas aussi, autant le dire, nous ne pensons pas que le projet de loi améliorera de manière profonde et significatif, la situation sur ces 2 points, une vraie réforme de l'orientation des jeunes devra apporter des réponses aux problèmes auxquels demain nos jeunes seront encore durement confrontés, des solutions existent pour aider nos jeunes à trouver une filière qui correspondent le plus à leur attitude, bien entendu, mais aussi aux perspectives d'emploi dans le marché du travail, mettre en place un système d'orientation qui commence et se continue jusqu'à la fin de la licence, donnant ainsi la possibilité un jeune en fonction de sa maturité et de sa capacité à se projeter dans l'avenir d'avoir différents tant d'orientation à condition bien entendu qu'il soit accompagné et durant toute cette période, voeux à nos jeunes un droit à l'erreur, en leur permettant de changer d'orientation en cours de ses années de lycée mais aussi au cours de son 1er cycle d'enseignement supérieur et enfin organiser demain le 1er site de manière plus souple dans un système modulaire capitaliser humble et semestriel. Ce n'est évidemment que dans le temps que nous apprécierons l'efficacité de la nouvelle plateforme d'affectation et d'orientation des étudiants tout d'abord en septembre prochain, en espérant que le sentiment d'incompréhension et d'injustice ressenti par certains étudiants et leurs familles, l'année dernière n'ait plus sa place cette année, mais au-delà, bien sûr, dans les années à venir, en espérant que la formation et l'accompagnement des bacheliers, et la réaffectation dans les différentes filières se fasse de manière plus pertinente et plus simple que par le passé un enseignement supérieur qui donne à chacun sa chance, c'est là le projet que nous centristes portant depuis toujours, c'est pourquoi nous voterons ce texte en attendant une réforme plus profonde de l'orientation, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe CRC. Madame

Madame la présidente, madame la mise, chers collègues, après les lois prix Pécresse de 2007 et Fioraso de 2013, le projet qui nous est proposé d'adopter définitivement ce soir constitue une étape décisive vers une autonomie toujours plus grande des universités en leur donnant la possibilité de sélectionner leurs étudiants votre gouvernement, Madame la Ministre, par la voix des députés de la République en marche, a finalement abandonné toutes précautions de langage, il et a trouvé facilement lors de la commission mixte paritaire de mardi dernier un accord global qui marque la victoire de la position défendue par le rapporteur du Sénat qui affirme sans tabou que la sélection est bénéfique et qu'elle est une chance pour tous ainsi cette loi que vous nous avez présentée comme technique et imposée par la nécessité de ne plus recourir à la pratique illégale du tirage au sort se dévoile enfin dans son véritable objectif de rupture radicale avec le principe général adopté à l'unanimité, il y a 50 ans dans ce même hémicycle de donner aux bacheliers, les mêmes droits de poursuivent leur formation dans l'enseignement supérieur, rompant avec cet idéal républicain que nous continuerons de défendre, vous organisez avec ce projet, la mise en concurrence des établissements déformation des diplômes et des étudiants vous donner aux universités la possibilité de s'inscrivent de s'investir comme des entreprises sur le marché de la connaissance et de l'éducation, les étapes suivantes de ce grand mouvement de marchandisation du savoir sont élevés à prévoir, c'est l'augmentation des droits d'inscription, le recrutement international des professeurs en dehors du cas de la fonction publique, l'utilisation généralisée de l'anglais pour l'enseignement et l'élaboration de filières d'excellence destinés aux étudiants étrangers, ces pistes sont déjà exploré par plusieurs universités et votre projet de loi leur donne une base légale pour poursuivre et accélérer ce développement, les vrais bénéficiaires de cette loi ne sont pas les étudiants, mais les établissements qui souhaitent aujourd'hui abandonné leurs obligations de service public pour s'engager dans la course à l'attractivité et tenter de gagner quelques places dans le classement de Shangai, considéré comme le parangon absolu du marché de l'éducation ainsi devenus les pépinières des premiers de cordée, ces établissements de prestige refoule auront vers des universités de relégation les indésirables, qui défendait en c'était 1000 cycle vos territoire ne doutez pas que cette course effrénée se fera aux dépens des petites universités que vous avez eu tant de mal à promouvoir et à défendre dans ce domaine aussi le ruissellement n'existe pas, nous avons tout à craindre d'un système universitaire à plusieurs vitesses et il n'est pas douteux que le renforcement des inégalités d'accès au savoir, aura des conséquences fâcheuses sur le niveau moyen de connaissance des futures classes d'âge nous savons toutes et tous dans cet hémicycle que les prochaines victimes de la rentrée de septembre, le 2018 seront les candidats qui choisissent définir généraliste l'université par défaut et que l'instauration de la sélection va les exclure définitivement de l'enseignement supérieur pour ces jeunes provenant principalement des filières technologiques et techniques, plusieurs groupes du Sénat avait proposé de réserver de nouvelles places ouvertes pour eux dans les IUT, toutes nos propositions en ce sens ont été rejetées, vous nous en avez en toute honnêteté, donner la raison essentielle, votre gouvernement, Madame la ministre ne souhaite pas ouvrir de nouvelles capacités d'accueil et fait le choix politique d'attendre l'inversion de la courbe démographique pour résorber le surplus de bacheliers indépendamment du bon fonctionnement ou non de la plateforme Parcoursup et quoi qu'il arrive, vous devrez, Madame la Ministre, en septembre 2018, assumer la responsabilité politique de l'éviction de tous ces jeunes, votre gouvernement il y a, ont décidé de ne pas attendent l'adoption définitive de la loi pour l'appliquer ces jeunes prennent peu à peu conscience, à la lecture des attendus de Parcoursup que leur origine sociale et le statut de leur laisser leur donne très peu d'chance d'accéder demain à l'enseignement supérieur, sans vouloir le reconnaître, nous savons très bien qu'il est très difficile de réussir la première année des études de santé sans recourir aux services supplémentaires d'officines privées pour un montant d'environ 4000 euros, le taux d'échec de 80 pourcent 1ère année Laura sur une clientèle captive et de substantiels bénéfices avec Parcoursup ces offres d'accompagnement privés viennent de connaître un développement spectaculaire, il est ainsi possible d'acheter pour environ 750 euros, un dossier tout prêt avec un Curriculum vitae parfaitement adapté aux attendus de la formation souhaité cette stratégie onéreuse sera d'autant plus efficaces que les dossiers de candidature seront nombreuses et exigeront des traitements informatisés en choisissant d'utiliser essentiellement les résultats des 2 premiers semestres de la classe de terminale pour choisir les candidats en réduisant les épreuves anonymes du bac que l'art du Baccalauréat, par le biais d'une réforme que vous gouvernement n'a pas de nier nous présenter, c'est une habitude, vous organisez une sélection sociale qui va avoir pour conséquence de renforcer l'escourgeon des élèves issus des milieux les plus populaires avec votre projet, Madame la Ministre, les universités ne sont plus les instruments d'une politique nationale mais des entreprises qui proposent des services à des des candidats qui doivent apporter les preuves sociale de leur capacité à correspondent à la cible de clientèle, ce modèle a opposée à ce modèle libéral notre idéal républicain de l'égalité des droits, d'accéder au savoir et à la connaissance. Merci bien, la parole est maintenant notre collègue Stéphane Piednoir pour le groupe, les républicains.

Madame la présidente, Madame le Ministre. Mais, chers collègues, nous arrivons donc à la dernière étape de l'examen de ce projet de loi avec la en plus sa dernière intervention, nous allons donc enfin donner un fondement légal à la procédure d'inscription des bacheliers dans un 1er cycle d'études supérieures. Comme je l'ai déjà souligné lors de la première lecture, le gouvernement a fixé un calendrier extrêmement contestable qui a court-circuiter l'action du groupe du Parlement, ce qui inquiète d'autant plus qu'il a volontiers recours au dispositif de procédures accélérées ou de procédures d'ordonnance ces derniers mois. Si l'on ajoute à cela le projet de réforme constitutionnelle, on peut s'interroger sur la place exacte que l'État souhaite accorder au Parlement. Pour revenir au sujet, il y a unanimité sur un point. Le dispositif APB devait être remplacés puisqu'il a mené à une situation de blocage dans les affectations et même de crise avec un recours illégal au tirage au sort l'an dernier. Je suis surpris, cependant, de certains choix qui ont été faits. Comment les établissements vont-ils pouvoir faire face à l'amoncellement des dossiers à examiner notamment du fait de l'absence de classement des dix voeu formulé par chaque candidat. Ne pas fixé 2 priorités dans les voeux permettra peut-être aux bacheliers de mûrir son choix quelques semaines supplémentaires, mais cette idée déconcerte par son évidentes difficultés de mise en oeuvre. On a parlé d'usine à gaz effectivement la tâche, les chefs d'établissement sort considérablement alourdi de cette réforme. Inévitablement, pour faire face au traitement des dossiers des algorithmes locaux verront le jour, sans contrôle national je ne suis pas certain que cela réponde entièrement aux recommandations de la CNIL. Le gouvernement réalise bien que la seule façon de traiter le problème du manque de place dans certaines filières et d'introduire une forme de sélection. En refusant de le faire, clairement, il multiplie les difficultés, obligeant les établissements à fixer des pré-requis attendus imposant des remises à niveau par des parcours personnalisés dont on ne sait ni comment ils seront financés, ni ce qu'ils apporteront vraiment. Notre rapporteur a recueilli l'avis de plusieurs universités qui estime que les nouveautés de la rentrée seront cosmétique et que dans certains cas, faute de moyens, les modules créés le seront en détruisant des modules existants. On peut également se demander à quelle date les établissements les moins demandées connaîtront leurs effectifs définitifs et comment la longueur de la procédure sera vécue par les jeunes concernés. Sans vouloir être d'un pessimisme primaire il me semble que les conditions sont loin d'être rassurés pour la rentrée universitaire 2018. Le Sénat a cependant pu apporter plusieurs améliorations du texte initial, parmi celles-ci, je soulignerai l'importance à mon sens de 2 mesures. Tout d'abord, concernant la proposition d'une formation aux jeunes n'ayant eu aucune, aucune n'ayant reçu par donc des réponses négatives, il est essentiel d'associer le directeur d'établissement à la décision du recteur. Notre rapporteur Jacques Grosperrin que je félicite au passage pour la qualité de son travail et sa recherche de consensus, a relevé le risque d'atteinte à l'autonomie des établissements et introduit en commission une obligation d'accord de l'établissement. La commission mixte paritaire est parvenu à une rédaction de compromis c'est vrai avec les députés, le recteur n'agira que dans la limite des capacités d'accueil et le directeur pourra proposer aux jeunes une autre formation ou bien un accompagnement préalables, il était en effet essentiel que les établissements et voix au chapitre. Autres points moins majeur que je souhaite évoquer la prise en compte des perspectives d'insertion professionnelle d'une formation lorsque le recteur détermine ses capacités d'accueil a été évoqué à l'instant. Le projet de loi ne traite pas le problème essentiel de la carte des formations. Je pense d'ailleurs qu'il aurait fallu prendre du recul et adopter une démarche globale, agir en amont sur l'adéquation des offres de formation à la réalité du marché du travail. L'accès à la saignements supérieur, n'en doutons pas une étape importante de formation intellectuelle pour construire son avenir personnel et professionnel. L'employabilité, l'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers actuels ou d'avenir sont aussi des objectifs en soi. Je considère qu'introduire la prise en compte par l'autorité académique de ces indicateurs pour augmenter les capacités d'accueil mais également éventuellement pour les réduire, est une mesure courageuse. Je me réjouis donc de cet apport du Sénat qui a fait l'objet de discussions vives parfois au sein de la commission mixte paritaire. Madame le Midi, ce projet de loi peut-être un point départ il est venu régler un problème ponctuel, celui de l'engorgement de certaines filières, mais pour combattre l'échec en 1er cycle universitaire, l'inégalité des chances et le chômage des jeunes, tout reste à faire, notre groupe espère donc que le gouvernement fera preuve prochainement d'ambition, je vous remercie. Merci, cher collègue, la discussion générale est donc Close, je rappelle qu'on application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat examine après l'Assemblée nationale, le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte et conformément à l'article 42 toujours alignés à 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de du dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, il y a-t-il des demandes d'explications de vote Monsieur David Assouline. Oui, tout ça pour ça, je je veux relever, comme beaucoup l'ont fait ici que sur la base du constat, parce que le conseil d'état parce que CNIL d'un système d'affectation qui n'était pas possible et pour préparer une rentrée, il fallait un nouveau système, on pouvait très bien, par décret, car ça ne relève pas de la loi décidée une période transitoire et une réflexion du Parlement de la société sur notre système universitaire, aboutissant à une vraie loi de réforme qui répondent, sujet que vous voulez traiter que vous affirmez vouloir traiter qui est celui de l'échec et de la sélection par l'échec de cette sélection sauvage vous y répondez et si vous n'est pas passé par décret, tout en prenant un peu en otage tout le monde puisque vous dites si on ne fait pas et si on ne vote pas cette loi, on est 800000 jeunes sans rien et l'avenir de nos jeunes est plus important que tout, sauf que par un système d'affectation pour répondre et corriger les fautes commises et en particulier la faute du tirage au sort que je reconnais tout à fait volontiers et sans problème, donc vous avez choisi autre chose si vous avez choisi de passer par la loi, c'est que vous lui donnez l'ambition de régler le problème de l'orientation et l'échec de la sélection par l'échec, vous institutionnaliser une forme de sélection et ce n'est pas mieux parce que vous verrez, et on fera les bilans ici au Parlement et on discutera que le nombre de jeunes qui vont rester sur le carreau, vous ne va pas tellement diminué les origines sociales de ce qu'ils vont réussir, ne vont pas tellement diminué, pourquoi, parce que si nous avions pris le temps, madame la ministre, de discuter, nous aurions pu traiter le problème plus globalement elles adossé à de, de, de programmation, c'est-à-dire à une discussion financière car l'orientation, le suivi plus personnalisé tous ces accompagnements que nous souhaitons tous, nécessite bien entendu beaucoup plus de moyens et nécessite un 1er cycle où on n'est pas entassés dans des amphithéâtres EDF les universités qu'on laisse dépérir, il faut beaucoup plus de moyens, si on n'est d'accord sur l'ambition, et donc je veux finir en disant que pire de n'avoir pas traité cela, vous avez décidé finalement de vous êtes d'accord avec la droite et cette loi, qui était la loi Duval est devenue la loi Duval Grosperrin, c'est ce que vous appelez le compromis mais en tous les cas, nous pensons que tout reste à faire et que cette loi va vraiment institutionnaliser une forme de sélection et ce n'est pas le chemin que doit prendre notre université. Merci, cher collègue, le j'mais aux voix l'ensemble du projet de loi à madame la présidente, monsieur, monsieur Pacaud Monsieur pas Kovanen à présent vous. Madame Morin Desailly vous préférez voilà. Oui, quelques mots suite à monsieur Assouline d'abord pour lui rappeler que notre ministre s'appelle Madame Vidal et non Madame Duval voilà, Madame la Ministre, je vous rends votre votre votre nom Talleyrand disait tout ce qui est excessif est un insignifiant, je suis obligé d'intervenir, monsieur Assouline quand je vous entends à nouveau dénoncé tout le travail que nous venons de faire cesser ces derniers jours par les 2 sélections sauvage de près de de précipitations, il y avait pas urgence on pouvait gérer les choses tranquillement, via un décret etc, moi je voudrais quand même rappeler que la la réalité dans laquelle nous nous trouvons, c'est tout de même bien la faillite du précédent gouvernement qui n'a pas su gérer la réalité d'abord de l'échec massif en en licence et l'inadéquation du d'un système de sélection qui s'est avérée illégal voilà, par la suite, donc je crois que il faudrait avoir su apporter des solutions à l'époque, prévoir la façon dont vous comptez vous y prendre pour permettre à nos jeunes, toujours plus nombreuses ces dernières années leur avoir permis de s'orienter de bien s'orienter et de construire leur parcours de de de réussite donc, où il y avait urgence il y a urgence, on ne peut pas laisser sur le bord du chemin des jeunes sont en train de passer leur Baccalauréat et qui s'inscrivent bien entendu dans des perspectives immédiates d'intégration vers l'enseignement supérieur, alors soyons tout de même positif il y du travail à faire, c'est certain, on l'a tous dit sur ces bons, bons, la minute, vous avez pris l'engagement, j'espère que vous reprenez aujourd'hui de revenir devant nous pour que nous puissions continuer à travailler et approfondir ces questions d'orientations qui vont revenir forcément dans le débat public à la faveur de la loi sur l'apprentissage, pour le reste vous avouerai qu'on a une petite frustration parce que l'on sait que la réforme la réflexion sur le lycée et l'évolution du Baccalauréat, ce sera d'or d'réglementaire, donc n'auront pas l'occasion vraiment d'en débattre pleinement comme nous faisons pour cette loi mais nous comptons sur vous pour être attentif aux travaux que nous continuerons à mener tout simplement dans le sens de l'intérêt général et l'approfondissement de ce sujet qui vous le savez nous tient particulièrement à coeur, nous l'avons démontré dans les années précédentes, donc voilà, ceci étant ayant été dit moi je voterai cette loi, je crois que le Sénat a été respectée dans son appréciation du sujet dans ses propositions, nous sommes parvenus à un texte d'équilibre à l'issu de la CMP, qui doit pouvoir donner à chacun la chance de trouver parler de réussite. Merci beaucoup, la parole est maintenant à monsieur Pacaud. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, monsieur le rapporteur, même si nous avons du nombre, renoncer à certains amendements certaines de nos volontés nos souhaits avec les différents amendements avec le partenariat fructueux entre députés et sénateurs, Madame le ministre et je tiens, moi aussi à saluer le travail particulièrement conciliant conciliateur fédérateur de Jacques Grosperrin donc la version finale du projet de loi constitue vraiment un 1er pas indispensable, indispensable vers une meilleure orientation ou au moins affectation pour les futurs bacheliers, un 1er pas indispensable pour sortir de l'ornière d'APB mais dans quelques mois, dans quelques mois, on pourra y voir, entre guillemets, plus clair sur les atouts mais aussi les limites du dispositif et puis comme l'a dit une dame Morin-Desailly, il va y avoir la réforme du Baccalauréat, la réforme du lycée, on y verra plus clair et moi je vous donne en fait rendez-vous je nous donne rendez-vous, je suis persuadé que dans quelques années, nous devrons revenir ici pour une vraie loi d'orientation et de réussite des étudiants alors serait à ce serait-ce sera une loi Vidal Grosperrin, je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'on y reviendra plus vite que prévu. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame il. Merci madame la présidente, moi je voulais intervenir pour parce que je me pose certaines questions, notamment quand on voit que tout ceci a été en fait générée par le taux d'échec en licence, or pour avoir été professeur toute ma toute une carrière, ce taux d'échec pour moi constitue quasiment un scandale et il impose de ne pas seulement mettre la faute aux étudiants, mais aussi se poser la question de l'enseignement lui-même pour avoir été professeur en collège et en lycée dès que nous avions des résultats au brevet et au bac qui ne différaient que de 1 pourcent par rapport aux moyennes qu'on avait obtenu l'rivière l'année précédente,

je pense que cela n'a même pas été envisagé ça me choque beaucoup, je trouve qu'on se trompe lorsqu'on veut classer les étudiants sort sans leur accorder la confiance, ce sont des être en devenir, c'est faire peu de cas de ce qu'ils sont, et de leur capacité, qui sont en général tellement supérieur à ce que, à ce qu'ils peuvent montrer donc voilà, moi je, je me demande si on est allé sur les bons sur le bon questionnement, voilà c'est tout, merci. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Sueur. Merci madame la la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voulais dire d'abord que ce débat illustres. Le fait que la procédure accélérée est extrêmement dommageable. Et sa généralisation, Madame la Ministre pose un véritable problème, en effet, pour ce qui est du rôle du recteur pour trouver in fine et une solution aux étudiants pour lesquels il n'y a pas de solution, vous avez proposé Madame le recteur un amendement devant le Sénat qui présenter un certain nombre de garanties. Or, après cet amendement on est arrivé tout de suite, et en CMP, il y a eu un compromis et ce compromis est fâcheux parce que Madame la Ministre, il est finalement quelque part en contradiction avec l'esprit de votre amendement, en effet, que dit le texte de la commission mixte paritaire, je vous assure, Madame la Ministre, c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues et cela a été très bien dit par Sylvie Robert par David Assouline avec mes collègues, moi je ne peux pas voter ce texte, c'est que la rédaction de la CMP, dit que le recteur peut trouver une solution qui doit trouver une solution quand la limite CD, capacité d'accueil qui ont été définies en amont, donc s'il y a un jeune qui est là, le recteur, plein de bonne volonté, dit mais je vais lui proposer. Une place mais la capacité d'accueil n'existe pas dans cette discipline dans cette, dans et par conséquent, Madame la Ministre, le texte telle qu'il était écrit ne peut absolument pas garantir que tout étudiant que tout jeune trouvent une solution, contrairement à l'exposé des motifs de votre projet de loi et là il y a une contradiction et je suis persuadé que une lecture complémentaire aurait peut-être permis d'avancer en tout cas je pense qu'il y a la problème parce qu'on va se retrouver dans des cas où des recteurs feront des propositions qui ne pourront pas être honoré et où par conséquent des jeunes seront exclus, or nous ne voulons pas que les jeunes soient exclus. Si chers collègues, est ce qu'il y a d'autres explications de vote non, et donc je vous propose de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans La rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur ces fameuses conclusions de la commission mixte paritaire, il va donc procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos Javid les secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin.

Voilà le résultat du scrutin numéro 63 sur l'ensemble du texte Compte-tenu de l'homme, l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs, ou groupe politique a notifié la présidence il y a eu 345 votants, 343 support phrase pour l'adoption 250 comptes 93, le Sénat a donc adopté ce texte le projet de loi est donc définitivement adopté, madame la ministre vous donne la parole. Merci infiniment madame la présidente, juste quelques mots : je voulais vraiment très sincèrement remercier la Haute Assemblée pour l'adoption définitive de ce texte, que dire que c'est un moment qui est évidemment extrêmement émouvant pour moi, mais je pense surtout que c'est un moment qui est extrêmement important pour les pour les jeunes qui vont passer le bac cette année, mais aussi pour ceux qui vont passer leur Baccalauréat dans les années à venir, je je remercie très sincèrement les sénatrices et les sénateurs de ne pas tous considéraient que venir de familles modestes interdit la réussite et que l'Intelligence ne s'évalue pas uniquement au niveau des comptes en banque et je pense que c'est très important que nous soyons en capacité d'aider l'ensemble des lycéens et l'ensemble des bacheliers à réussir dans l'enseignement supérieur, parce que tous ceux qui ont leur place à condition d'y a 3 compagnies et c'est l'objet de cette loi, je vous remercie très sincèrement. Merci, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant de lever la séance, je vous donner lecture de lors du jour du mardi 20 février 2018 de 15 heures à 16 heures, explication de vote des groupes sur le projet de loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à 16 heures 30 scrutin public solennelle en salle des conférences sur le projet de loi organique à 16 heures 30 proclamation du résultat du scrutin public solennel ne à ses heures 45, les questions d'actualité au gouvernement. Et à 17 heures 45 débat sur les conclusions du rapport d'information femmes et agriculture pour l'égalité dans les territoires, à 21 heures 30 débat sur l'avenir de l'audiovisuel public, chers collègues, la séance est levée.